La séance est reprise, nous reprenons la discussion du projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la Covid 19 dans la discussion des articles, nous sommes parvenus aux explications de vote sur les amendements identiques numéro 7 30 rectifié bis 38 rectifié bis et 62 au sein de l'article de et nous avons les explications de vote qui ont été déjà demandé Monsieur Chassaing. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, sur effectivement les articles que vous avez cité, madame la présidente, mais aussi sur l'article trente-huit j'ai pas pu le faire tout à l'heure, donc je ne vois pas dans la demande de tester à 12 ans de discrimination ou d'hostilité vis-à-vis des jeunes, les jeunes ont très bien compris que l'efficacité pour se préserver de la contagion qui peut être massive et Ambos lisez l'hôpital et l'économie, il y a certains virus, donc comme le centaure qui paraît très agressif, beaucoup de descendants. Il faut tester isolé tracé vacciner, vacciner pour éviter les formes graves et diminuer la contagion, ce ne sont pas les tests qui coûtent cher, mais les hospitalisations en soins critiques réa 9 malades sur 10 en soins critiques RN il mation ne sont pas vaccinés, ce sont des faits et ce ne sont pas des accidents de la route transformée en Covid comme c'est écrit dans l'amendement de 38, allez voir les médecins urgentistes et en réanimation, 9 sur 10 ne sont pas vaccinés en réa, c'est aussi le cas à Tulle et à Brives, que j'ai rencontrés, et donc il y a pas beaucoup de personnes âgées en fait mais des gens qui n'ont pas été vaccinés et je voudrais vous dire aussi que, avant la vaccination, l'entrée en virus Nepad était un véritable cauchemar pour les médecins, bien sûr les les directeurs le soignants les soignants et les familles, il faut donc tester les jeunes à partir de 12 ans et la Papou lation pompe pas déborder en hôpital et conserver l'activité économique, merci. Merci madame Müller Bronn. Merci madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre, chers collègues, alors je reviens sur cette idée de ne de, de faire un test aux enfants à partir de 12 ans on aurait aimé et beaucoup de parents, beaucoup de structures scolaires, périscolaires de grands-parents auraient aimé éviter que les enfants entre 12 et 18 ans lorsqu'ils ne sont pas majeurs soit soumis, encore une fois, à des mesures qui qui sont oppressante, qui sont, qui ne sont pas favorables à leur je voudrais juste dire que le Sars Covid de. Est une zoonose et donc touche plus de 40 espèces animales y compris les animaux domestiques, alors si nous voulons nous mettre sous cloche que le virus très dangereux n'entre pas par les adultes n'entre pas dans notre pays par les enfants, que faisons-nous avec les animaux, les animaux domestiques, vous n'êtes pas sans savoir que le hamster importer du Pays-Bas a été la source établi d'une Rodrigue recrudescence épidémique à Hong-Kong, une étude publiée dans le lent cette a mis en évidence la diffusion du du virus par les frontières internationales via le commerce des animaux et on sait que les containers transportent des animaux de compagnie, malgré donc les passes et malgré la vaccination humaine, nous n'y arriverons pas, comment voulez-vous faire est-ce qu'on doit créer un test aussi pour que les animaux n'apporte pas le virus très dangereux sur le territoire national. Merci Monsieur Bénard Roche. C'était juste une question, au fait que j'avais, vous savez que je nous avons déposé un amendement dans ce sens là, donc, pour faire en sorte que la vacciner le Pass voyage ne soit demandé qu'à partir de 18 ans, et j'ai entendu une argumentation me semble-t-il, dans la bouche de, de, de Monsieur le Ministre, faisant état en fait du du toutes sortes de taux de contagiosité ou du nord de contagiosité qui étaient liés ou ou qui étaient dues à des personnes entre 10 et 19 ans, alors j'ai peut-être mal compris, d'abord, je voulais avoir peut-être cette précision est-ce que est-ce que qu'est-ce que c'est que ce taux est où via-t-il et deuxièmement si c'est entre 10 et 19 ans

Merci madame la présidente, il y a quelque chose de juste dans ce que dit Madame Noël notre collègue Noël c'est que il y a aucun dispositif qui permet, à coup sûr d'arrêter un virus à l'entrée, sur un territoire est-ce qu'on tire de ce constat. La décision de ne rien faire. Ben c'est ce que vous proposez et je suis encore une fois étonné que sur les mêmes bancs ce qui réclamaient la fermeture totale des frontières, ce virus qui vient de l'étranger, bla aujourd'hui adopte la position inverse, c'est-à-dire on ne fait rien. La question qui se pose à nous, c'est la question de la maille du filet. Pour essayer de retarder l'entrée éventuelle d'un variant dangereux parce qu'on est quand même dans l'hypothétique Il y a une question qui est de trancher et oui, ça pourrait être, disons, ça pourrait être cinq ans, ça pourrait donc la la décision, elle est politique, on peut décider de ne rien faire et de dire ses 18 ans même ou 20 ans ou 30 ans. Et là, il a été dit, il est proposé 12 ans. C'est une maille qui me paraît raisonnable est-ce que ça a des effets problématique j'ai entendu invoquer des trous psychologique, alors c'est une question sérieuse, ce qui a été l'impact notamment des confinements de la privation d'activités sociales pour les enfants et pour les jeunes pendant la première phase de la pandémie. Mais pardon, ne transposons pas ça sur le fait de réaliser un test parce qu'on va prendre l'avion pour aller à New York pour revenir de d'un département d'outre-mer, non franchement invoquer la un trouble psychique, psychologique chez les enfants ou une mesure disproportionnée, j'ai entendu aussi le thème me paraît pas très recevable, donc ce qui est proposé là l'âge de 12 ans et raisonnable, oui je discute si vous aviez déposé un amendement disant je ne sais pas pourquoi pas mais en tout état de cause, je ne vois pas d'arguments sérieux pour voter ces amendements qui consisterait à relâcher les mailles du filet. Merci, cher collègue Madame Gouache avant. Madame la présidente merci pourquoi 12 ans en fait moi, ça me paraît, je suis pas une grande spécialiste mais un peu au doigt mouillé, on parle de justement Monsieur Jomier viens de dire 10 ans ben tiens, pourquoi pas neuf pourquoi pas 13 pourquoi pas 14, enfin il y a un moment oui on me souffle pourquoi pas 2 ans, mais il y a un moment, je crois que bornons-nous à ce qui avait été voté, ce qui avait été proposé à l'Assemblée nationale, pourquoi faire plus strict, plus invasifs parce que certains enfants à 12 ans vivent très mal le test PCR dans le nez, hein, je peux vous le dire autant peut être à dix-sept dix-huit ans ça passe mieux, ah oui, oui, évidemment, vous n'avez que des enfants parfaits, j'imagine qu'il supporte tout en attendant moi j'ai des retours de personnes qui me disent : oh la la les tests vous savez sont pas fait tout le temps de la même manière, ils sont pas toujours fait de manière très douce et et parfois, c'est un petit peu difficile à vivre pour les enfants, donc voilà, c'est juste une question moi je pose la question : pourquoi 12 ans pourquoi revenir sur une disposition qui finalement était très logique parce que 18 ans, c'est finalement la majorité et je trouve que c'est assez logique, personnellement, je voterai ces amendements. Merci. Alors, je vais mettre aux voix, donc ces quatre amendements identiques, donc le sept, le 30 rectifié le 38 rectifié le 62 qui ont reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ne sont pas adopté 2 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune le 55 présenté par Monsieur Bonnecarrere. vous avez tous écouter la présentation de notre rapporteur, l'article 2 est divisée en en 2 parties, une partie, une qui concerne les transports internationaux, une partie de qui concerne les transports entre la Corse, les outre-mer les outre-mer et la métropole, la partie une les transports internationaux et dans l'esprit de notre rapporteur, traité, sur la base de l'apparition de variants, le gouvernement pourrait, en cas d'apparition d'un variant quelque part dans le monde reprend des dispositions dites de filtrage pour reprendre la formulation qui a été utilisé tout à l'heure pour la relation avec l'outre-mer et la Corse, la logique est différente et elle s'appuie exclusivement sur l'idée de ne pas créer de situations surcharge hospitalière outre-mer cette seconde logique a conduit notre rapporteur à une rédaction dans lequel il prévoit que seuls les trajets entre la métropole et Outre-mer ou la Corse pourrait faire l'objet de mesures préventives de la part du gouvernement, c'est rationnel, puisque c'est la logique à partir de laquelle il a construite sa rédaction, le seul problème que nous n'avons pas vu immédiatement, c'est que chacun le sait, vous avez par exemple, les mouvements de population réguliers entre le Brésil et la Guyane, vous pouvez en avoir entre Les Hauts plateaux africains et Mayotte, entre autres exemples, si demain vous avez un virus qui un variant qui apparaît au Brésil, vous pourrez assurer une filtration entre récifs ou Rio de Janeiro et Paris, mais vous ne pourrez pas le faire entre la Guyane et Paris la rédaction, cet amendement vise à permettre de corriger ce trou dans le filet pour reprendre une formulation qui a été utilisé également dans la situation du trajet dans le sens retour j'ajoute que la commission des lois, il y un regard favorable sur cet amendement dont la rédaction est alignée sur celle de mes collègues qui vont intervenir leur rédaction, ils ont été plus complète, merci. Merci l'amendement 65 donc identiques, présentée par Monsieur Mohamed Soilihi. merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les motifs de notre amendement viennent d'être exprimés avec clarté par notre collègue Philippe Bonnecarrère je veux rappeler que cet amendement est en cohérence avec l'article approuvé en commission un amendement de protection du territoire contre les variants qui sont susceptibles de circuler à l'étranger dans des pays limitrophes, faut-il rappeler le cheminement des variants d'état et Delta, lesquels ont eu un rôle actif dans de précédentes vagues, je veux bien insister ici sur les points suivants tout d'abord, au terme de cet amendement des conditions et critères d'application du certificat au déplacement depuis les outre-mer sont resserrés par rapport au droit en vigueur ensuite l'amendement conserve plusieurs modifications intervenues lors des débats à l'Assemblée nationale puis lors de l'examen en commission au Sénat, s'agissant de l'application du certificat pour les déplacements à destination des outre-mer notre amendement prévoit d'ailleurs lui-même la consultation des exécutifs locaux et des parlementaires, des collectivités d'outre-mer concernés un un mot d'une application du certificat pour les déplacements depuis les outre-mer, enfin c'est ces dispositions consistent seulement dans une faculté que le gouvernement ne pourrait mettre en oeuvre que jusqu'au 31 janvier 2000 23 au plus tard dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid 19 de manière strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu et qu'il devra cesser d'appliquer sans délai lorsqu'elle n'est plus nécessaire, je cite ici la loi je merci. Ainsi l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Avis favorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Madame la présidente, monsieur le le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs. Le caractère insulaire de la plupart des Outre-mer et la proximité de pays étrangers, connaissant une situation sanitaire très diverses qui ont effectivement donné lieu à l'apparition de nouveaux variants, Brésil, Afrique du Sud, nécessite de permettre l'application de la mesure aux voyageurs en provenance des outre-mer à destination de l'Hexagone pour éviter une plus forte diffusion du virus, le caractère très touristique de ces tueries Touaregs et les brassages particuliers auxquels ils sont exposés sont également à prendre en compte à cet égard. En outre, la symétrie que vous souhaitez instaurer entre l'Hexagone et les Outre-Mer existe dans notre droit depuis l'introduction du Pass Frontières sans que cela et soulever et soulever de difficultés particulières auparavant. Votre amendement maintient maintient ainsi déséquilibre existant. Et on sait que la mesure est utile vers l'Hexagone comme entre territoires ultramarins pour limiter la diffusion de nouveaux variants a paru à l'étranger qui entreraient sur le territoire par les Outre-mer dans tous les cas, je rappelle que vous ne votez là qu'une habilitation instaurer le Pass variant lors des déplacements depuis les outre-mer à destination de l'Hexagone ne sera mis en oeuvre par la première ministre que si nécessaire, enfin l'amendement prévoit la consultation des exécutifs et parlementaires concernés avant toute application du dispositif garantissant une décision concertée avec les populations ultramarines, ce que je ne peux qu'approuver, pour ces raisons avis favorable. Merci, alors oui, me sert nous. Merci madame la présidente, aux Français d'outre- mer c'est con, vous partez de la Bretagne pour la à Paris, on peut vous demander un Pass, c'est exactement le même message que vous venez d'envoyer ces cons vous venez d'un territoire ultramarin de Saint-Pierre-et-Miquelon pour aller vers l'Hexagone on peut exiger, à un moment donné la preuve que vous ne soyez pas atteints de Covid alors vous me direz, c'est une possibilité, monsieur le ministre et je vous ai entendu effectivement moi je parle du symbole et du message qu'on envoie au territoire si certains ici n'ont pas encore compris que le résultat des élections, on a connu cette année avait été impacté et heurté complètement par la manière dont la crise sanitaire avait été sur certaines mesures qui n'ont pas été prises écoutez par les exécutifs locaux, merci monsieur le rapporteur, d'avoir intégré les exécutifs au niveau de l'avis donné par le représentant de l'État sur les mesures envisagées, je pense qu'on n'a pas encore compris le message qui est envoyé à nos d'ultramarins et c'est vrai que le vrai message intégré dans le texte de la commission, c'est une protection parce que le vrai sujet, pour nous, c'est la pénétration du virus sur notre territoire. Pour éviter le risque de saturation et c'est pas l'inverse, même si, effectivement, Monsieur le Ministre, a du brassage de chacun dans nos bassins géographiques, c'est pas vraiment le sujet d'ailleurs, il suffit d'observer le décalage dans le temps de la crise sanitaire en outre-mer par rapport à l'Hexagone, je pense que c'est simplement faire preuve de pragmatisme et moi sincèrement et je l'ai dit à mes collègues, je m'opposerai à ces deux amendements qui sont de mon point de vue un mauvais message envoyé aux outre-mer on voyait à tous les Français, parce que quand vous partez d'un vol direct ultramarins vers l'Hexagone, on peut vous demander une preuve de la même manière que celle qu'on peut exiger à l'entrée sur le territoire français, mais on est en France. Et peut-être qu'il faut encore le rappeler, visiblement et ça n'est, semble-t-il, pas tout à fait clair je vous remercie. Merci Monsieur Lurel. Madame la présidente, monsieur le milicien collègue je partage totalement l'avis de mon collègue Arnaud mais totalement parce que le message, il a envoyé là, c'est de dire que si 2 mais il devait y avoir une circulation, encore plus intensive du virus, il ne peut être importé des outre-mer. On est en train de le créer là une sorte de frontière virtuelle que je ne comprends pas, et je peux entendre, voir, comprendre le sens de l'amendement, mais je ne peux pas l'approuver, de dire que, en fait, pour résumer ça il y a asymétrie ce que l'on demande au départ de la métropole, hé bien, on va l'exiger aussi au départ de de aujourd'hui vous Jean oh, ça, ça n'existe pas aujourd'hui, vous êtes en train de changer un système qui fonctionne depuis pratiquement 2 ans, je ne comprends pas quel est le motif même leur apporte qui pourtant fin et subtil juriste n'a pas osé demandé ça et c'est vous qui demandez ça en ostracisant davantage mon compte, j'aime pas mais que je vais utiliser les autres mais je vais voter contre ces deux amendements.

mes chers collègues, tout ce qui est excessif est vain, je viens d'entendre parler d'ostracisation, je viens d'entendre parler d'un message qui ne serait pas passé souvenez-vous lorsque cette pandémie a commencé, nous étions les premiers à notre mère a demandé la protection de nos territoires, a demander de la solidarité, cet amendement, c'est de la solidarité parce que nous ne pouvons pas nous contenter de demander de la solidarité et qui y des mesures de protection et de contrôle, au départ de la métropole et à partir de nos territoires, nous en laver les mains, alors que nous savons que des variants comme le 501 qui est né en Afrique du Sud, hé bien, a fini par gagner le monde entier, l'Afrique du Sud, c'est un territoire qui se trouvent pas loin de Mayotte pour partir de l'Afrique du Sud à Mayotte, il y a un moyen très simple, on va aux Comores et puis des Comores à Mayotte, vous savez c'est une passoire, nous passons notre temps à le dire ici de la même manière du Brésil en Guyane et ce qu'il faudrait taire cette situation juste parce qu'on n'est pas en train de parler d'immigration clandestine, hé bien moi, je suis désolé, c'est une solidarité que je dois à mes collègues de l'Hexagone n'importe qui à n'importe quel moment peut passer de l'Afrique du Sud à Mayotte, du jour au lendemain, et c'est d'ailleurs comme ça que le le le variant 500 et a commencé à inquiéter parce que connu en Afrique du Sud, hé bien, on a détecté aux Comores. Donc, moi, c'est, c'est la raison d'être de cette de sa main, cet amendement, je pourrais dire : on est protégé en partant de de l'Hexagone, on est tranquille, mais je pense que le variant peut partir aussi de nos territoires vers l'Hexagone. Merci, cher collègue Je voudrais dire tout simplement qu'il faudrait qu'on soit à un moment donné cohérent. Tantôt, on parle de continuité territoriale. Alors, il faudrait qu'on sache ce qu'on veut vraiment merci. Merci. Alors, je vais mettre aux voix ces deux amendements donc 55 et 65 qui ont reçu un avis favorable de la commission et du gouvernement qui est pour.

écoutez on va vous demander un assis debout, je suis désolé, ça va vous faire bouger vous endormir et moi. Alors. Qui est pour.

qui est contre.

il s'abstient. Ils sont adoptés. Je vous remercie. Cet amendement faisant l'objet d'une discussion commune le quarante Si madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons déposé cet amendement parce que nous avons été stupéfaits du texte que le rapporteur a fait adopter par la commission des lois, texte qui supprime l'obligation qui fait une croix sur le Pass sanitaire pour appuyer la sécurité sanitaire du pays exclusivement sur les tests PCR. Que recherche nous que cherche-t-on s'il y a la menace d'un nouveau variant de, de protéger au maximum le territoire. Nous savons depuis 2 ans, qu'aucune mesure de protection aux frontières n'est totalement étanche au mieux on freine et on fera une suffisamment pour mieux connaître le variant. Et on a vu comment on pouvait y parvenir avec la combinaison de tests PCR de la vaccination ou des certificat de rétablissement pourquoi après 2 ans ton au fameux test PCR d'il y a 2 ans, monsieur le rapporteur, c'est assez problématique c'est aussi assez problématique par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur le respect du droit européen le certificat Vert, Union européenne, il dit bien mobilité pour ceux qui ont un test PCR ou bien un certificat de rétablissement ou bien un certificat de vaccination, donc c'est assez étonnant que maintenant vous nous fassiez le contraire, j'ajoute que aucun les,

j'ajoute aussi que toute mesure qui qui freine et s'il y a des tests, les tests PCR ne sont en rien une garantie si a un variant qui galope, parce que si il y a un variant qui galopent et qui menace, vous demandez aux gens de faire des tests voulait relancer la relâcher dans la nature pendant 48h avant qu'ils voyagent, ils peuvent chopé le le le variant et après vous les ferai venir de toute façon c'est pas certain et en plus, parmi les nouveaux variants, il peut y en avoir qui ne sont pas visibles par l'État, tests, merci, donc ça fait que nous souhaitons, nous souhaitons rétablir le texte telle qu'il l'était auparavant comme un certain nombre de amendements de de nos collègues. Merci monsieur le comte l'amendement numéro 19 Madame Müller Bronn. Oui. Merci madame la présidente, alors c'est un un amendement qui prévoit que la durée de validité des examens de dépistage virologique soit inscrite dans la loi est ainsi conforme au certificat européen ceci est indispensable pour éviter que le gouvernement n'impose par décret une durée réduite à 24 heures comme il l'a fait le 25 novembre dernier ce qui avait mis d'ailleurs en difficulté de nombreux Français, tant dans leurs déplacements, ainsi que dans leur vie quotidienne et ce, sans preuve scientifique de son efficacité, merci. Merci alors 4 amendements identiques, puisque le 67. Es retiré,

pourquoi, je vais essayer de développer 2 autres arguments le le 1er c'est que la mesure contraignante de présenter un test de dépistage négatif et que celui-ci nécessiterait en fait parallèlement la gratuité de ces tests pour garantir à tous citoyens ultramarins Corse et citoyens de l'Hexagone, la libre-circulation sur notre territoire, or il est nul, envisager de rock gratuit ces tests de dépistage pour les personnes non vaccinées à moins que monsieur le ministre, ici présent ne soit venu faire des annonces en ce sens, il nous le dira. le dira. 2ème argument aussi, c'est celui de la cohérence de nos politiques, la position du rapporteur Philippe Bas de resterait de l'accès des déplacements à la seule condition de présentation de tests de dépistage semble ajoutée nous semble-t-il, de la confusion au message de prévention et de politique vaccinale adressés aux Français depuis ces dernières années, ces derniers ont joué le jeu puisque au 17 juillet 2000 va de 80 pour 100 des Français avaient bénéficié d'un schéma vaccinal complet, ils sortent donc dès lors très curieux d'envoyer un message politique contraire en leur imposant Maitland à nouveau la réalisation de tests pour leurs déplacements, j'oserais dire d'ailleurs, je voudrais rappeler que nous avions été les premiers ici même à ouvrir le débat sur la 3e dose a fait faire de schéma vaccinal complet, une véritable protection pour la population, je rappellerai qu'il n'est pas justifiée sur le plan sanitaire d'exclure le certificat de rétablissement de la Covid 19 des modifie des modalités de certificat sanitaire de voyage dès lors qu'il est établi que ces personnes récemment contaminées guéri ne présente pas de risque de recontamination, dans l'immédiat, je ne vous ferai pas la fraude ressortir les argumentations du ministre de la Santé précédent qui lui-même étaient réticents à la présentation d'une preuve de non-contamination par test, les restrictions de la libertés fondamentales et autres la bande la liberté d'aller et venir, doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et doivent être également nécessaire et proportionnée, les auteurs du présent amendement ne considère pas que ces conditions soient réunies en l'espèce, sans la modification que nous proposons, ainsi qu'un certain nombre de nos collègues.

donc si vous voulez, c'est expliqué tout à l'heure par l'amendement socialiste le présent amendement a donc pour objet de rétablir la faculté pour les voyageurs de présenter l'un des 3 documents que constituait le passe sanitaire, c'est-à-dire effectivement le taf statut vaccinal ou certificat de rétablissement alors effectivement le le l'argument selon lequel seul un test négatif pour empêcher la propagation du virus, c'est efficace, mais le vaccin et aussi efficace, mais pas à 100 % parce que si on veut faire un test, il faudrait le refaire après une quarantaine, mais bon, par ailleurs, il apparaît primordial de continuer à encourager la population à se faire vacciner, à l'heure où la quatrième doses de vaccin est ouverte aux personnes les plus vulnérables, enfin et surtout, ça a été dit, cette disposition ne pas conforme à l'esprit du du règlement européen selon la l'article 3 du point cette dispose ainsi que la délivrance des certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner discrimination fondée sur la possession d'une catégorie spécifique de certificat visées à l'article 5, certificat de vaccination de tests certificat de rétablissement, donc c'était dans un but de cohérence qui paraissait important puisque si vous voulez, ça paraît à la lettre à la rencontre de ce qui se passe au niveau européen, il paraît important de maintenir la possibilité pour les voyageurs de présenter l'un des 3 documents constituant le certificat Covid numérique de l'UE. Merci le 54, monsieur Bonnecarrere. Oui, nous sommes là sur le seul sujet qui fâche : notre groupe et que nous n'avions pas du tout, imaginez que nous n'avions pas vu arriver si les amendements que nous présentons ne sont pas adoptés, cela veut dire que demain en situation de crise. Seul peut être rétabli l'obligation passer un certificat de ne de se faire tester pour pouvoir se déplacer. Regardons demain, regardons le passé, si on regarde, demain, à partir du moment où il n'y a plus aucune disposition qui donnent une pertinence, une conséquence au fait d'être vacciné, cela veut dire que vous avez officiellement considéré que le certificat de vaccination n'a aucun intérêt et derrière nos concitoyens ne peuvent que comprendre que s'il certifie la carte de vaccination n'a pas d'intérêt, la vaccination n'a pas le même d'intérêt, c'est toute la contradiction pour demain, tous dit sur les différentes bancs que l'on avait besoin de la vaccination, plus que jamais pour assurer la protection collective, nos concitoyens, et là on adopterait une mesure si vous ne nous suivait pas qui va à l'encontre de la vaccination et si maintenant vous regardez le passé et je fais quand même un appel à la cohérence des positions qui ont été défendue par Philippe Bas et par le président Retailleau pour de votre groupe depuis le début, vous avez pris une logique à laquelle il faut rendre hommage, de vouloir protéger les populations, vous avez donc voter les différents textes, malgré les difficultés que ça représentait pour chacun de nous sur les passes sanitaires si demain officiellement on dit que le certificat de vaccination n'a pas le même intérêt que le test, cela revient à dire que pendant 2 ans nous avons imposé à nos concitoyens, des choses qui ne serait pas justifié, vous imaginez la suite, les anti-vont sans gros frais dans cette brève dans cette brèche et dire que l'ensemble du dispositif que nous avons les gens et les autres, adopté au fur et à mesure des des lois étaient inadaptées conquérir nous raconter des histoires à nos consommateurs, je ne crois pas raisonnable. L'amendement 56 n'est pas défendu alors je demande sur ces amendements, l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente, je voudrais mettre à part l'amendement numéro 19 rectifié vous apporter la réponse de la Commission sur cet amendement, immédiatement, c'est un amendement qui vise à ce que la durée de validité du test pour pouvoir embarquer dans un pays qui serait affectée par un variant du Covid extrêmement dangereux qui serait soudainement apparu ne puisse pas être de moins de 72 heures Madame mais nous a expliqué tout à l'heure que, effectivement, quand on a exigé des tests, il est arrivé que le gouvernement exige un test de 24 heures cette ah bon droit et pour de bonnes raisons, que le gouvernement l'avait fait le ministre lui dira mieux que moi, mais c'est tout simple : si la nature même de ce variant en fait qu'un test de plus de 24 heures n'a pas de valeur parce que le la, la, la contamination peut fort bien se faire dans ce cas il faut laisser la liberté au gouvernement en fonction du variant il faut toujours pouvoir s'adapter à la réalité et donc notre avis est défavorable, pour des raisons qui ne sont pas de principe mais qui sont de pratiques alors maintenant nous avons un certain nombre d'amendements qui visent tous à dire que face à une situation tout à fait exceptionnel. Et fort improbable de d'émergence dans un pays donné, d'un variant extrêmement dangereux qui exigerait qu'on prenne des mesures protectrices pour les Français, à l'intérieur de nos frontières, on puisse demander avant l'embarquement, non pas simplement un test négatif. Mais une vaccination à jour ou un certificat de rétablissement, là aussi, les choses ont changé depuis un an, rester crispé sur des positions qui était juste, il y a un an et qui serait devenue mauvaise serait de la mauvaise législation. Aujourd'hui, quels sont les changements, ben ils sont multiples. Le virus est plus viral, le virus est moins dangereux. Et surtout, le vaccin. Ne protège actuellement ne fait barrière à la contamination actuellement que dans un tiers des cas. Il reste une protection nécessaire et je crois qu'il faut le rappeler pour chaque individu, surtout s'il est vulnérable. Mais il ne fait pas barrage. Dans plus d'un tiers des cas à la contamination, vous le savez tous par conséquent, dire que si il y a. Un nouveau variant. Du Covid. Qui surgit quelque part si ce variant est très dangereux et si pour protéger la France, on demande simplement un vaccin jour alors que déjà avec les variants actuels. Dans des 2 tiers des cas, le vaccin ne fait pas barrage à la contamination et donc à la con, tu agis auditer de la personne atteinte, hé bien, c'est très simple, on rate notre cible, on ne protège plus, alors bien sûr, de tout le monde le sait bien c'est médical, c'est pas un problème politique, il n'y a pas de sécurité absolue évidemment le test peut rater sa cible dans certains cas, évidemment, si le test est trop ancien, le virus peut faire son oeuvre sur l'organisme du sujet qui s'est fait tester mais bien sûr, c'est vrai, mais au fond, face au choix qu'on va avoir pour protéger dans une situation exceptionnelle et fort improbable le territoire national, le choix qu'on va avoir, c'est un choix pratique vous voulez être efficace, vous demandez le test, le test est inconfortable, c'est plus facile parce que la plupart des gens sont vaccinés, c'est plus facile de demander le vaccin, et bien je ne vous propose pas la solution de facilité, sachant que maintenant il n'y a plus de passe vaccinal, il n'a plus de passes sanitaires il n'y a plus aucune mesure de contrainte que ça ne changera pas la vie des gens c'est pour au fond : avoir un filet de sécurité qui n'est appelé à jouer que de manière tout à fait exceptionnelle mais tant qu'à faire que de mettre ce filet de sécurité autant qu'il soit efficace, mes chers collègues, et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment en toute sincérité et en toute humilité devant les lacunes des connaissances que nous pouvons avoir dans ce domaine, particulièrement quand, comme c'est mon cas, on n'est pas scientifique, on n'est pas médecin, on n'est pas biologiste et au fond, nous n'avons pas l'être pour être bon législateur nous devons simplement utiliser correctement les informations qui sont à notre disposition sans fantasmer sur les messages qu'impliquerait éventuellement les dispositions comprend ce que nous devons faire, c'est voter pour des dispositions utiles et non pas voté pour conjurer de mauvaise interprétation de la loi, soyons très concrets, précis, pragmatique et efficace, c'est la raison pour laquelle je vous propose, en ce qui me concerne, de rejeter ces amendements identiques pour des raisons de fond qui me paraissent très importantes et qui sont de traiter correctement une situation particulière dont j'espère comme vous, qu'elle n'arrivera jamais. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs. Nos amendements tendent à réintroduire le justificatif de statut vaccinal et le certificat de rétablissement parmi les éléments du Pass variant et du Pass, outre-mer. Comme vous l'indiquez la vaccination, une infection à la Covid 19 réduits pendant un temps significativement le risque de survenue de formes graves. Mais également. Elles réduisent le risque de transmission à autrui. Quand bien même elle ne l'empêche pas totalement. Ainsi exiger la présentation d'un certificat de rétablissement ou un justificatif de statut vaccinal continue à faire sens. Sens médicalement. Essence dans un message de clarté, de santé publique. Les personnes disposant de ces documents présentent moins de risques d'hospitalisation et de surcharge du système de santé monsieur le Leconte. Vous proposez toutefois que ces documents ne puisse être exigé que de manière alternative et non cumulatives. à l'égard des voyageurs en provenance des pays classés en zone rouge, c'est-à-dire ces pays où il y a une très forte circulation active de la Covid 19 ou un nouveau variant dangereux, il est nécessaire d'être en mesure de demander un vaccin ou un certificat de rétablissement. Et un test, pas seulement l'un ou l'autre. Médicalement je ne peux pas dire autre chose. Le régime actuel en vigueur de combinaison d'épreuves est applicable depuis plus d'un an sans difficulté. Il n'est pas nécessaire, ni souhaitable de réduire le Champ des possibles sur ce point, alors que l'épidémie nous a déjà réservé de mauvaises surprises dans le passé et nous impose l'humilité. Cette combinaison sera décidée au cas par cas en fonction du risque. C'est pour cela que je m'engage devant vous. à ce que si votre haute assemblée retenait le principe d'une consultation obligatoire sur la mise en oeuvre du Pass Frontières l'organisme scientifique, appelés à se prononcer, s'exprime aussi sur la combinaison en cause afin de garantir publiquement que celle qui sera retenue par décret l'aura été en fonction d'éléments objectifs, transparents et médicaux. J'entends vos arguments, monsieur le rapporteur, mais en tant que médecin, je ne peux qu'être favorable aux amendements qui maintiennent le droit en vigueur et vous invite monsieur le comte à retirer le vôtre à leur profit. Madame Müller Bronn votre amendement, quant à lui, prévoit que l'examen de dépistage virologique doit avoir été réalisée au maximum 72 heures auparavant. Comme vous le savez, la durée de validité des tests dépend des connaissances scientifiques, en particulier en cas d'apparition de nouveaux variants et de la situation sanitaire. Elle Elle tient compte aussi des pratiques de nos voisins, afin d'assurer la plus grande cohérence possible dans des espaces de libre-circulation comme l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle cette durée déterminée par voie réglementaire, après avis de la Haute autorité de santé cette manière de procéder d'éclairage scientifique en temps réel et une capacité d'ajustement permanente par décret, il n'apparaît pas souhaitable de rigidifier les choses aujourd'hui au niveau de la loi. Par ailleurs le règlement européen 2021 953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ne précise pas que la durée de validité des examens de dépistage virologique doit être fixé à 72 heures, il se borne à définir le cadre juridique du certificat Covid numérique, de l'Union européenne, qui doit être acceptée par l'ensemble des États, sans préciser les durées de validité du résultat d'examen de dépistage virologique la certificat de rétablissement et d'un justificatif de statut vaccinal pour ces raisons avis défavorable. Merci madame la présidente, Le rapporteur nous a invité à ne pas avoir un raisonnement figé moi je partage totalement cette façon de penser. Hé bien, si on ne ne veut pas avoir un raisonnement figé en toute humilité toute sincérité, on doit dire que personne d'entre nous n'est capable de dire si le prochain variant qui surviendra peut-être le de 75. Le meilleur outil, ce sera d'avoir un certificat de vaccination ou de faire un test PCR pour se garantir que la personne ne va pas amener le variant. Or, par votre position, monsieur le rapporteur, vous nous privez automatiquement de ces outils, vous n'en conserver qu'un seul parce que vous présupposé que parce que, actuellement, c'est le meilleur outil, ce sera le meilleur outil dans 2 ou 3 mois, mais nous nous réunirons pas à nouveau dans 2 ou 3 mois, et donc il est plus sage de laisser ouvert la possibilité de ces différents outils. Ceci dit, nous avons entendu ce qu'a exprimé le ministre et donc la nécessité de ne pas non plus fermer dans un choix binaire, donc nous allons adapter notre position pour que le meilleur texte soit adopté dans quelques instants, à cet égard, et je voudrais dire aussi ne se rapporteur que en figeant en fermant comme ça la situation autour de la seule pratique du test PCR, vous sortez le vaccin. Symboliquement, du statut d'outils nous permettant de nous protéger, or, si c'est un outil, un parfait sur la transmission, bien sûr, il ne réduit que partiellement le risque de transmission, c'est tout de même un outil qui a une certaine efficacité et là vous envoyer un message peut être à votre corps défendant, mais à ceux qui luttent contre le vaccin comme vous envoyez un vous enverrai un peu plus tard dans la discussion, un autre message et nous ne partageons pas ses messages, il ne s'non son ni juste sur un plan scientifique ni adapté sur un plan politique. Merci monsieur le comte. Qui n'est pas à sa place. à partir du mot, je comprends que Monsieur Bonnecarrere maintiendra son son amendement, nous retirons notre amendement au profit de celui de Monsieur Bonnecarrere, nous appelons tous ceux qui sont attachés à la sécurité sanitaire des Français a envoyé de la part du sénat un message sur la question de l'efficacité des vaccins, a voté un amendement qui, effectivement, assure la sécurité sanitaire des Français dans un contexte qui est toujours. Pas certain, nous sommes très étonnés que en 6 mois, monsieur le rapporteur, soit passé de d'une personne qui nous fait voter le passe vaccinal à une personne qui ne veut même plus maître le vaccin comme un élément de contrôle message vis-à-vis de l'efficacité du vaccin ne nous semble pas très opportun, il est important de maintenir l'ensemble des dispositifs et j'entends monsieur le Ministre de choses si nous tenions initialement à ce que ce soit l'un ou l'autre ou le 3ème, je vous indiquer la raison dans un certain nombre de pays, les tests PCR coûte très cher, jusqu'à 150 euros par personne pour une famille avec 2 enfants, ça peut être un blocage à un retour en France, c'est-à-dire à l'incapacité d'arriver dans un pays où vous avez une capacité de soins, la 2ème chose c'est lorsque vous êtes français et que vous vivez à l'étranger et que vous n'avez pas le bon schéma vaccinal si on exige une combinaison des 2, alors il y a un problème. Donc, nous retirons cet amendement au profit de celui de monsieur Bonnecarrere, mais nous vous demandons à trouver des dispositifs qui n'exclut aucun Français qui vit à l'étranger, de la capacité de revenir en France, lorsqu'il se trouve en danger dans une zone qui est menacé par un variant particulièrement grave. Merci Monsieur Bénard Roche. de notre groupe et aussi celui des indépendants et je rajouterai d'ailleurs que les 2 amendements qui ont été retirés au moment de la séance, celui qui était présenté par Monsieur Alain Richard et Mohamed il pour des pays et celui qui devait a défendu, il me semble pour RDSE était également les mêmes donc je pense réellement c'est aussi l'avis du ministre donc je pense réellement, monsieur le rapporteur, que c'est essentiel pour faire en sorte que cet article 2 soit voté par l'ensemble des bancs de cette assemblée, ce qui serait quand même une bonne chose que vous puissiez accepté de donner un avis favorable à cet ensemble d'amendements qui viennent de pratiquement tous les groupes qui sont représentés ici. Il avait pas, il avait pas Merci madame la présidente, je pense que la l'intervention et la déclaration du ministre Brown nous éclaire ce soir sur le sens qu'il est, être porté par la haute assemblée sur une discussion importante, je vous remercie, Monsieur le Ministre, puisque par votre intervention, vous nous amenez en ce qui nous concerne, a retiré l'amendement numéro 40 sur lequel nous étions prêts à à envisager un scrutin public et nous nous rabattent on mais au meilleur sens du terme sur les amendements présentés par les autres groupes parce que, effectivement, vous nous avez rappelé le le bon chemin à suivre, je ne vais pas être très agréable, monsieur le rapporteur et vous voudrez même en excuser par avance. Il y a beaucoup d'incendies de forêt en ce pays et ce soir vous avez manif manipulé ou manifester une forme de d'enfumage généralisé vis-à-vis de plusieurs groupes de notre assemblée, je le dis ici très simplement. La raison qui est la vôtre, que vous avez présenté de manière la plus scientifique possible n'est pas que scientifique, elle est aussi liée à une situation politique qui vous lie à un autre groupe à l'Assemblée nationale, et je ne souhaite pas, je ne souhaite pas que les débats politiques qui sont ceux de la haute assemblée soit liée finalement à des contraintes et des considérations qui sont celles et ceux de la majorité LR ici présente, je le dis très simplement, parce que sur un sujet aussi important sur lequel nous nous sommes tous battus à savoir favoriser, encourager et presque pour ce qui nous concerne, obligé à la vaccination, nous soyons obligés de faire un retour en arrière, ce qui est tout à fait inacceptable au regard des enjeux de santé publique dans notre pays, donc je le dis très simplement, nous voterons par un scrutin public favorablement aux amendements apportés par nos collègues, notamment monsieur Bonnecarrere parce que nous estimons que c'est le bien de la nation qui est en cause, monsieur le rapporteur. Merci monsieur le questeur sueur. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, chers collègues, si nous sommes nombreux à intervenir, c'est pas ce que nous voyons bien qu'il y a là un événement d'une certaine gravité, en cet instant au Sénat. Parce que il y a 48 heures, monsieur le rapporteur, vous étiez tout à fait favorable à ce qu'il y a eu les 3 modalités le vaccin le test et le certificat de rétablissement et puis votre pensée a évolué et il est difficile de ne pas penser en effet que la situation complexe qui est celle de l'Assemblée nationale peut conduire certains et après tout. Il y aurait une logique à imaginer qu'il faudrait que nos débats ici soit guidé par le fait de favoriser telle ou telle vote de tels ou tels groupes à l'Assemblée nationale, mais moi je dis que c'est grave parce que la question est de savoir ce qu'on pense, ce qui nous paraît juste et vrai et je crois que le bicamérisme suppose que chaque assemblée se détermine par rapport à elles-mêmes et puis après on verra, il existe une commission mixte paritaire et donc il est très important, me semble-t-il, alors que nous sommes très nombreux je pense au combat de nos amis d'outre-mer. Très difficile. Pour défendre le vaccin face à des oppositions irrationnel. Nous avons défendu le vaccin. Que aujourd'hui nous ne revenions pas en arrière pour des questions d'opportunité, je crois que ce qui se passe à l'assemblée se passe à l'Assemblée, mais ne doit pas d'éteindre. Sur ce que nous allons faire au Sénat en toute indépendance, c'est comme ça que doit fonctionner la république. Madame la présidente. J'ai demandé à mon groupe de retirer l'amendement que nous présentions et qui était dans le sens de la convergence d'autres amendements et celui du gouvernement. Je l'ai fait pour une raison principale qui est le raisonnement praticien défendue par Philippe Bas. Nous devrons de toute façon le gouvernement en fonction lorsque une nouvelle situation de circulation inquiétante se développera devra utiliser les moyens les plus applicable et plus pratique pour traiter cette nouvelle situation de circulation virale. Le vaccin. Sera moins adapté. à cette situation et d'en faire donc une une preuve en quelque sorte, concurrente du test viral virologique ne nous semble pas ne me semble pas au moment où on parle comme une solution adaptée, j'ai entendu l'argument du ministre et j'ai été frappé que par l'engouement du gouvernement, ils disent en tant que médecin, je ne peux pas prendre une autre position, j'entends tout à fait je respecte cette approche, mais en l'occurrence, il s'agit de faire marcher, un système de contrôle public dans une situation de crise et il me semble que il vaut mieux se tenir à l'utilisation du test qui décrit la situation et qui permet d'identifier la situation de circulation la plus récente la plus réelle, alors que l'utilisation du vaccin ou d'ailleurs du certificat de rétablissement qui date de 3 mois ou 6 mois serait un signe trompeur, il me semble donc que c'est un motif déterminant en tout cas c'est celui qui m'a déterminé à choisir de ne pas suivre cette logique-là, et se on peut s'adresser des procès politiques faut on avec plus ou moins d'élégance, mais il se trouve que, en l'occurrence la simple réalité conduit à cette solution. Merci monsieur ou père. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le président Richard parlé avec beaucoup de sagesse, on parle des tests, on parle des vaccins et je suis très heureux que le le rapporteur ben dis implicitement que le meilleur passe sanitaire, c'est par le contrôle des tests. Revenons au vaccin, moi ce que j'ai appris en tant que praticien c'est qu'un vaccin efficace, il est fait avec la souche la plus récente et on a prouvé que le vaccin que le le le virus Omicron le variant Omicron ne réagissait pas aux vaccins et j'ai peur que dans l'avenir les variants futurs ne réagissent pas,

merci madame veut rien. Merci madame la présidente, alors quel est l'objectif de se protéger, très clairement, outre le fait de ne pas contaminer, c'est surtout de ne pas engorger nos hôpitaux, on le sait, or qu'est ce qui permet le mieux de ne pas engorger nos hôpitaux et ça aussi on le sait, c'est le vaccin parce qu'effectivement ça n'empêche pas d'attraper la maladie, ça empêche juste d'aller en réanimation d'aller aux urgences et d'aller engorger nos hôpitaux, c'est bien ça l'objectif du vaccin, maintenant je me mets dans la le cas d'une famille qui va voyager, il va aller passer ses vacances à l'étranger dans un pays. Quel qu'il soit, peut être même la Suisse un pays frontaliers qui tout d'un coup devient rouge, on ne sait pas pourquoi, voilà, il y a et donc pour pouvoir revenir alors peut être que la Suisse, pas le meilleur exemple parce que je pense qu'on trouve assez facilement ou aller faire un test PCR, mais malgré tout, pour les frontaliers qui vont devoir faire un test PCR à chaque fois qu'ils vont devoir aller travailler tous les 48 heures, vous vous souvenez de cela, tout ce qui n'est pas à faire maintenant qu'on est vacciné et que on peut voyager grâce à ce vaccin, hé bien il va falloir le faire et alors si on est dans un pays plus éloignés, on est en vacances avec sa famille et on doit trouver comment avant son départ en avion aller faire son test PCR le payer éventuellement très cher et imaginez un des membres de la famille française qui est en vacances quelque part qui doit revenir et un des membres, l'un des enfants est positif, vous faites quoi vous laissez-vous rester toute la famille vous annulez tous vos billets d'avion vous quinze jours et vous rentrez pas chez vous, c'est bien ce qui se passe et donc, si l'objectif c'est d'éviter d'emmerder les Français puisque ça été reciter peut être que de fait de garder 3 possibilités, c'est-à-dire la guérison, le vaccin ou le test PCR, ce qui n'oblige donc aucunement à la vaccination et permet aussi de s'en sortir probablement ça laisse beaucoup plus de souplesse pour voyager pour les Français comme pour les étrangers d'ailleurs.

de savoir que si au bout de deux mois trois mois telle ou telle mesure était la plus efficace, je rappelle simplement que le 2ème alinéa de l'article prévoit que si de ce positif et mis en oeuvre par le gouvernement, s'il doit être prolongé au bout d'un mois, il doit repasser par le Parlement, donc en réalité votre inquiétude s'éteint toute seule puisque, si au bout d'un mois, on ne sait pas si c'est le meilleur dispositif qui fonctionne, on pourra revoter. Merci Monsieur Hervé. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voulais insister sur le fait que, au 31 juillet au soir et ça n'est pas le sujet de ce soir, mais il va se passer quelque chose, c'est que le Pass vaccinal et le Pass sanitaire vont mourir de leur belle mort donc, mes chers collègues, si on parle de l'incitation à la vaccination, au travers de mesures comme le passe vaccinal au Pass sanitaire, cet argument ne tient pas puisque ces dispositifs n'existeront plus, là on parle d'un dispositif très particulier qui consiste pour l'essentiel ah imposées pour le trafic aérien. La réalisation d'un test PCR pour l'intégralité des passagers, on pense dans les exemples qu'on peut citer quand même souvent, je l'ai moi-même vécu, ma chère collègue, je pourrais vous donner l'exemple, mais quand par exemple il a un de de territoires d'outre-mer où le test PCR était obligatoire, vous vous êtes positif vacciné ou pas, vous n'embarquez pas. Moi, le 31 décembre j'ai fait un test à la Réunion, j'étais vacciné trois fois j'étais positif, j'ai, je, je, je, je n'ai pas remarqué et je me suis mis en quarantaine, donc si on veut avoir une garantie certaines, indépendamment du statut vaccinal, je répète, j'ai été vacciné trois fois sûrement une garantie certaine que aucun passager n'embarque en ayant le la Covid on teste tout l'avion, on teste tout l'avion on force tout l'avion à un test PCR et on exclut forcément les autres dispositifs le certificat de rétablissement ou le certificat de vaccination qui ne sont pas en mesure d'apporter la preuve que la personne n'est pas porteuse du virus, c'est la raison pour laquelle mes chers collègues, je ne voterai aucun de ces amendements et je suis très attaché à la rédaction proposée par Philippe Bas en tant que vacciner et au au titre aussi la défense des libertés publiques. Merci Monsieur Joyandet. merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans un moment de notre travail de législateur ici au Sénat, je ne parle pas de l'Assemblée nationale, mais ici au Sénat, justement, on est en train de légiférer en tirant des plans sur la comète et dans un moment, je reviens sur les propos de notre rapporteur, qui se place dans le cas d'une nouvelle épidémie très forte subite et cetera et nous ne savons rien de ce qui va se passer à ce moment-là, et moi je veux prendre date pour vous dire que, quoi, quel que soit le texte qu'on va voter ce soir il sera inapplicable et si le si, si toutefois la circonstance venait à surgir telle qu'elle est envisagée par notre ami Philippe, je pense que la meilleure solution c'est de revenir devant le Parlement, de regarder la situation de quoi il s'agit, nouveau variant pas nouveau variant les tests marche, il marche pas aujourd'hui, tout est dans la nature, moi je vais aggraver notre cas dans les constats parce que on dit on teste l'avion tout l'avion, bon c'est très bien qu'aujourd'hui vous avez des gens qui ont Covid symptomatique, j'ai beaucoup de témoignages vécus qui sont négatifs pendant quatre jours et qui sont positifs au bout du 5ème jour alors que ça fait six jours qu'ils sont contaminants donc mes chers collègues, nous ne savons rien de ce qui va se passer, et là on est chacun donne là chacun donne sa sa certitude, moi ce que je suggère, pour être sûr d'avoir juste que c'est juste d'avoir juste c'est de rejeter cet article-là et puis revenir devant le Parlement, quand on aura des vrais éléments factuels, on nous dira : où sont les virus, quels sont leur intensité de quoi on a besoin tout ce qui est proposé sur tous les bancs ne concerne absolument pas, absolument pas la situation future on essaie depuis une situation actuelle de déduire ce qu'on va faire dans un moment où on sait pas ce qu'on aura à faire, c'est quand même un peu ubuesque et ça, c'est pas l'Assemblée nationale, j'ai été élu Benjamin de cette maison en 95 j'ai vécu des bons moments, mais le moment qu'on est en train de vivre ce soir mais je ai. Merci, franchement, je n'ai pas vécu beaucoup et donc je veux vraiment prendre date le rapporteur, mais c'est ce qui passe, la parole est même présidente mais pas pris beaucoup la parole, je veux simplement dire que

c'est moi qui décide ici c'est moi qui préside donc quand je dis qu'on qu'on arrête, c'est terminé, vous êtes trop nombreux à prendre la parole, je ne peux pas laisser merci merci beaucoup madame la madame la présidente, je crois que nous sommes à un moment important dans les différents échanges et je crois que c'est bien, c'est très bien qu'on officiant de cette manière-là parce qu'en fait nous nous rendons compte que la situation, elle est devenue complexe, mais une chose est sûre, le vaccin a ses limites, la cinétique vaccinal, j'en ai parlé il y a quelques temps ici même la cinétique vaccinal, hé bien elle est à court terme. D'une part, d'autre part, le vaccin n'est pas efficace tous les mutants sud il n'est pas efficace il était peut être efficace pour certains, certains, mais avec tous les variants qu'on a toutes les mutations qu'on en aura jamais un vaccin efficace et c'est la raison pour laquelle, moi je suis très favorable au fait qu'il y ait des tests, le test permet le test qui sont PC, on peut être antigénique permettra de d'avoir à un moment donné, la situation de la personne et ce que nous avons pas fait et que le gouvernement a refusé il y a quelques mois, c'est la sérologie, on aurait pu voir justement le statut sérologique des gens, le taux d'anticorps qu'ils ont, on dit que ce n'est pas efficace, mais ce ne serait, elle est un indicateur, ce serait sans doute un indicateur important, donc je crois qu'au moment où nous nous sommes là, maintenant, c'est intéressant, mais nous avons tous et toutes, pratiquement je dirais était vacciné une fois deux fois trois fois probablement peut-être 4 ou 5 fois, tout simplement parce que nous n'avons pas de réaction liée au type de virus en fonction de la période, donc il est vrai que nous aurons probablement un virus beaucoup plus plus important qu'il y aura peut-être de faire des formes très grave, mais aujourd'hui je crois que faire des tests, faire des tests, il faut la privilégier alors pour les personnes déjà vaccinées, je ne dis pas que parce que des personnes ne seraient pas vaccinés aujourd'hui qu'il y aurait à être offensés, non, je crois que nous sommes tous et toutes, conscient que beaucoup d'entre nous ont été vacciné une fois, 2 fois, 3 fois et que régulièrement nous voyons dans nos bancs des personnes qui ne sont pas là parce qu'ils ont le virus parce qu'ils ont pas forcément le même virus alors tout simplement pour vous dire que nous devons faire preuve d'humilité mais d'axer notre action sur la prévention, merci. Merci madame autant. Merci madame la présidente, je vais faire une une explication de vote assez courte déjà priori moi je reste favorable au à la proposition de dire qu'on peut avoir le test, le vaccin ou le certificat de de guérison, quelque chose qui est scientifiquement et médicalement reconnue, donc on ne va pas réinventer ici les études et refaire, refaire de la médecine dans cet hémicycle, moi ce que je crois et ce que je ressens, c'est qu'on est sur une période de compromis aujourd'hui dans cet hémicycle faut faut se le dire, qu'on essaye de chercher la voie de passage la plus adaptée pour que le texte soit équilibré puisse arriver en son terme, donc moi je pense que si cette solution-là et la bonne ben il faut y aller, c'est pas la peine de cumuler le peut-être le Pass vaccinal enfin le pas, on est plus sur un Pass sanitaire parce que quelqu'un dit qu'il allait tomber effectivement, mais dans le passe sanitaire, il y a à la fois le vaccin à la fois le test et à la fois le le certificat de de guérison par contre, l'un n'exclut pas l'autre et je ne vois pas en quoi mettre le vaccin sauf si. C'est un irritant qui devient une limite rouge donc mettre en en le maire et le vaccin n'enlève rien à ceux qui veulent pas le faire, et du coup peuvent quand même faire leur tests hein, je ne vois pas ce que l'un empêche de l'eau, donc je serais favorable à ces amendements. Merci. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 19 de Madame Müller, Bronn, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est donc pas adoptée, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par les groupes, les républicains et socialistes sur les amendements identiques 6 36 et cinquante-quatre et je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable et l'avis du gouvernement est favorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter Le scrutin clos. Merci,

et notifié à la présidence Nombre de votants : 343 Nombre de suffrages exprimés 263 pour l'adoption 236 contre 27 Le Sénat a adopté. Alors 2 amendements feu. Dans l'objet d'une discussion commune le numéro 31 de madame Vogel. Merci madame la présidente, donc, dans une ordonnance du 18 août 2020, le Conseil d'État avait rappelé que le droit pour un ressortissant français établis à l'étranger d'entrée sur le territoire national était une liberté fondamentale, partant de là, cet amendement a vocation, essayer de respecter cette ordonnance du Conseil d'État et de concilier la nécessaire protection sanitaire avec la protection de la liberté fondamentale des Français établis hors de France, il y a donc 2 dispositions : l'une qui est simplement d'inscrire clairement dans la loi que les exigences ne saurait interdire le retour sur le territoire national, d'un ou d'une ressortissante française et la 2ème chose c'est d'inscrire la possibilité que les tests soient effectués à l'arrivée pour les Français qui sont à l'étranger, je voudrais préciser tout de suite que non ça n'implique pas, sauf si évidemment quand le gouvernement applique cette loi, il fait n'importe quoi, ce que je ne saurais croire que des Français prennent l'avion ou le train, en étant positif et en contaminant de tout le monde parce qu'ils feraient leur tests à l'arrivée ça n'implique pas forcément ça cette disposition, c'est juste pour offrir une base légale au gouvernement qui permettent d'autoriser des tests à l'arrivée pour les cas où ce soit indispensable au respect de l'ordonnance du Conseil d'État est possible dans le respect des exigences sanitaires appropriées, je vous rappelle par ailleurs que les personnes qui sont dans cette situation sont souvent vaccinés mais peuvent être dans des situations le schéma vaccinal du pays dans lequel ils vivent ne permet pas de respecter le le schéma vaccinal français parce qu'ils ont pas accès aux mêmes vaccins et une possibilité bien sûr pour éviter qu'ils soient discriminés serait de rendre les tests pour rembourser au gratuit, si le gouvernement fait ça il aura pas besoin d'appliquer cette cette possibilité, mais voilà, c'est simplement. Une possibilité, une base légale pour éviter les discriminations. je vais, je vais vous demander juste parler un tout petit peu moins fort pour qu'on puisse laisser les nos collègues défendent leurs amendements, s'il vous plaît. Merci. Alors le numéro 64 Madame Vargas oui allant dans le même sens. Cet amendement vise à aménager les modalités, l'usage du certificat sanitaire de voyage afin de ne pas pénaliser les ressortissants français de l'étranger qui souhaitent se rendre sur le territoire sur notre territoire national. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. la commission des lois a émis un avis défavorable, malheureusement sur son amendement parce que, une fois que les personnes sont arrivées sur le territoire national, si dans une situation où il s'agit d'un virus d'un variant du virus très dangereux si leur test fait uniquement à l'arrivée sur le territoire national est négatif, il faut encore décider de ce qu'on va faire de ces personnes et ça va être la quarantaine, je ne suis pas sûr que ce soit mieux pour elle d'avoir une quarantaine à l'arrivée sur le territoire national que de retarder un petit peu son voyage donc pour ces raisons assez pratiques et tout en voyant bien votre intention positive à l'égard des voyageurs, nous pensons que ça n'est pas leur intérêt en réalité d'adopter ce genre de dispositif, la vie est donc défavorable et il est aussi défavorable sur l'amendement numéro 60 IV parce que, en réalité, il il s'agit pas d'interdire le retour de qui que ce soit sur le territoire national mais ça d'attente, juste un peu que les conditions soient redevenues favorables pour que la protection de nos concitoyens sur le territoire national soit assurée, donc si vous acceptez de de retirer votre moment, je crois que ce serait préférable, sinon l'avis de la commission a été défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs. Les amendements tendent à prévoir à des dispositifs spécifiques pour les Français de l'étranger afin qu'ils ne puissent se voir refuser le retour en France. Madame Vogel vous proposer, ainsi qu'un test de dépistage leur soit proposé à leur arrivée sur le territoire pourtant permettre aux Français de l'étranger, de réaliser un test à leur arrivée sur le territoire national viderait le Pass variant de sa substance, en effet, comme cela a été rappelé, vise à freiner l'arrivée sur le territoire national de ce nouveau variant, or cet amendement permettrait aux Français de l'étranger alors qu'ils viennent d'un pays ou un nouveau variant circulent et sont éventuellement porteurs de celui-ci d'être en contact avec d'autres voyageurs durant leur trajet en avion en train. Et serait à leur présence sur le territoire, le risque de contamination, être avérée, sauf comme ça l'a été dit à mettre tout le monde en quarantaine, madame la sénatrice témoin d'observer que le Pass, outre-mer n'est applicable qu'aux trajet entre l'Hexagone et les collectivités ultramarines et ne peut avoir pour effet d'interdire un retour sur le territoire national, d'un ressortissant français. De manière générale le droit fondamental de tout Français de rejoindre le territoire national se concilie avec l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique, la jurisprudence admet que des restrictions peuvent être apportées si le bénéfice pour la protection de la santé publique excède l'atteinte portée à ce droit fondamental l'émergence éventuelle d'un nouveau variant avec des caractéristiques inconnu à l'étranger, justifie de protéger le territoire national, en instaurant un Pass variant qui s'appliquerait temporairement aux Français résidant à l'étranger, en revanche, comme vous le savez, il a été jugé qu'qui ne peut être imposée de motif impérieux aux nationaux pour revenir sur le territoire et le projet de loi ne revient pas sur ce point, pour ces raisons avis défavorable. Merci monsieur Chantrel pour explication de vote. ça n'est pas anodin du tout ces deux amendements parce qu'il y a eu un précédent assez grave, de par je dirais votre gouvernement c'était dans c'était en janvier 2021, mais bon, c'est le même gouvernement, il y a eu quelques petits changements c'est dans la continuité, il y a eu un précédent très grave à la fin du mois de janvier 2021 où il y a un décret qui a été pris, qui a exigé des motifs impérieux pour nos propres ressortissants qui n'était pas en France, c'est-à-dire que ce jour là, le gouvernement a décidé de faire le tri. Auprès de ses propres ressortissants. Ah, l'opposition même des conventions qui ont été rappelés justement européenne de sauvegarde des droits de l'homme des principes qui énumère clairement le principe du droit fondamental d'un ressortissant de pouvoir rentrer et sortir de son pays, et quand je vous dis que c'est un assez un précédent grave, ça a été d'ailleurs on a mené la fronde au Conseil d'État qui a cassé cassé ce 2 pourquoi c'est un précédent grave parce qu'il y a des personnes encore moins bien intentionnés que vous, qui sont d'ailleurs pas forcément dans cette assemblée, mais dans l'autre, qui feront également le tri entre nos ressortissants sur d'autres critères. Et c'est en ça. Que, en tant que législateurs, nous devons sécuriser pour que ce genre de choses n'ait plus lieu et en votant pour cet amendement, c'est ce que nous ferons. Monsieur le comte. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, si les Français sont dans un territoire où ils sont en danger, justement parce qu'il a ce variant et que vous ne permettait pas assez français de rentrer parce qu'il n'y a pas la possibilité de faire le test, nous avons connu ça il y a quelques années, qu'est-ce que vous leur répondez rester là où vous êtes, ce n'est pas notre problème qu'est-ce que vous leur répondez : c'est bien pour ça que nous déposons cet amendement. Merci, monsieur le Ministre. et comme je l'ai déjà dit auprès de l'Assemblée, je m'engage, au cas par cas par des mesures de gestion à régler ce genre de problème pour récupérer nos ressortissants qui serait coincé entre guillemets à l'étranger, dans ce cadre de situation. merci. Je vais mettre aux voix l'amendement 31 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour.

nos, nos compatriotes qui sont établis hors de France, qui n'ont pas forcément justement la possibilité d'avoir accès vaccin ou à, ou à des tests à des dépistages et que justement en cas d'entrée en vigueur du du dispositif prévu au 1er alinéa de l'article 2 privent de leur droit fondamental que que je vous ai exposées précédemment cet cet amendement, il prévoit justement que le gouvernement puisse établir après concertation avec les conseillers des Français de l'étranger, puisqu'en plus on a la chance d'avoir des élus à travers le monde qui vivent dans des, dans les pays concernés, donc qui ont une expertise qui ont la possibilité justement de dire les faits dans leur pays, il y a des accès ou non au vaccin, s'il y a des accès ou non aux tests PCR et de de permettre justement à travers cette cette concertation, d'avoir une liste des pays où le présent décret finalement ne ne s'appliquerait pas afin de de permettre, chose sur laquelle vous vous êtes engagé justement, Monsieur le Ministre, de permettre à nos ressortissants d'accéder au territoire national. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Il est défavorable, madame la présidente. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre,

Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune d'amendements 51 Monsieur La présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, donc si vous voulez, c'est simplement que le délai d'un mois, nous sommes trop court entraîne une sollicitation du Parlement qui n'est, semble pas justifié cet amendement vise à supprimer ce délai permet au gouvernement de prendre des mesures de prévention jusqu'au 31 juillet 23. Merci l'amendement 53 même qui autant c'est c'est un amendement de repli qui prolonge au-delà de moi. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame le président, cela mérite qu'on s'y arrête un instant, c'est vraiment la marque de fabrique du Sénat que de ne pas vouloir donner des pouvoirs exceptionnels au gouvernement sans exercer son contrôle et c'était une règle que nous avons toujours appliquée, on dit au gouvernement s'il y a urgence, vous pouvez restreindre les libertés dans un but d'intérêt général, mais pas plus d'un mois sans un vote du Parlement, donc du coup ces deux amendements qui l'un l'un vise à retirer l'intervention du Parlement et l'autre à allonger le délai d'un mois à 2 mois ce que nous n'avions pas fait jusqu'à présent, on te fait l'objet d'un avis défavorable de notre commission. Merci, monsieur le rapporteur, l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, concernant la demande de m'en 51, monsieur le sénateur votre amendement vise à supprimer la clause de revoyure parlementaire un mois qui a été adopté par la commission une clause de revoyure reprend un mécanisme propre à la prorogation de de régimes d'exception, la prorogation de l'état d'urgence, fondée sur la loi du 11 avril 1955 ou de la, de 12 jours et de l'état d'urgence sanitaire, au-delà d'un mois, nécessitant une autorisation du Parlement à défaut le droit commun est rétabli le présent projet de loi acte la fin des régimes d'exception d'état d'urgence sanitaire et de la gestion de la sortie de crise sanitaire désormais le droit commun redevient la norme. Ce dispositif est uniquement transitoire, il n'est applicable que jusqu'au 31 janvier 2023 et tous les dispositifs actuels de contrôle parlementaire renforcé des décisions que l'exécutif est amené à prendre en ce domaine sont maintenus par le présent projet de loi sans qu'il soit besoin de prévoir dans voter une nouvelle au bout d'un mois. Cela étant, le gouvernement tant la volonté de votre commission de prévoir cette clause de rendez-vous, j'aurai l'occasion de préciser que le délai d'un mois est en tout état de cause, trop court et je vais le faire mais sur le principe même de cette nouvelle clause de rendez-vous qui augure a peut-être, d'un 4ème projet de loi d'urgence sanitaire, le gouvernement s'en remet à la sagesse de votre haute assemblée. Concernant l'amendement 53. L'amendement vise à allonger à 2 mois le délai de la clause de revoyure parlementaire lorsqu'un nouveau variant de la Covid est détecté des études, des études pardon scientifiques prennent davantage qu'un mois pour identifier ces mutations la transmissibilité sa gravité son échappement à l'immunité conférée par les vaccins ou une infection à un variant préexistants. Face à un nouveau variant, dont les caractéristiques ne sont par définition pas encore connue, afin de ne pas exposer la population française, un danger, il est préférable. D'immédiatement réagir ainsi le variant Delta, dont les études sont en ont ensuite démontré qu'il présente une transmissibilité moindres mais une gravité accrue a été d'accepter en octobre 2020, selon l'OMS, toutefois, il n'a été classé comme variant préoccupant que le 11 mai 2021. On ne disposant que d'un seul, moi, il est très peu probable que les études scientifiques puissent établir suffisamment la dangerosité ou non d'un nouveau variant de la Covid 19. le dispositif ne pourra certainement pas être prolongé ce délai trop bref risque de nous amener à initier un grand nombre de projets de loi qui n'aboutiront pas, ce qui ne servirait pas l'objectif poursuivi pour sévère pour ces raisons, pardon : avis favorable à cet allongement du délai de la clause de rendez-vous. Merci, alors je vais mettre aux voix l'amendement donc 51 rectifié, qui a reçu un avis défavorable de la commission, a un avis de sagesse du gouvernement. Monsieur Chassaing, vous voulez prendre la parole à vous retirer votre amendement très bien merci, Alors donc je mets aux voix l'amendement 43, qui a reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour,

Merci madame la présidente, la commission des lois, suivant l'excellent travail de son excellent rapporteur a réintroduit un amendement LR adopté à l'Assemblée nationale avant que l'article de ne soit supprimé cette disposition prévoit la consultation des élus des collectivités d'outre-mer exécutifs locaux et parlementaires en cas de rétablissement du Pass sanitaire pour s'y rendre, il m'a paru cohérent que cette consultation des élus soient étendus à ceux des Français établis hors de France, alors que nous discutons de la possibilité de réinstaurer le passe sanitaire aux frontières pour venir en France, en effet, les élus des Français de l'étranger, dont une partie est représenté à l'Assemblée des Français l'étranger peuvent apporter des informations pertinentes sur l'état sanitaire des pays dans lesquels ils vivent comme alerter sur les capacités de tests, ils peuvent utilement éclairer la décision du gouvernement, c'est le sens de l'amendement que je vous propose. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Je comprends très bien de de l'amendement de nos collègues et ils ont sûrement raison sur un point, c'est que les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger ont des choses à dire, mais mettez-vous de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du côté des autorités sanitaires, un variant extrêmement dangereux apparaît dans un pays, croyez-vous réellement possible de réunir à Paris l'Assemblée des Français de l'étranger pour prendre des mesures urgentes, hé bien non, c'est impossible, c'est pratiquement impossible de faire ceci induirait des délais de consultation qui empêcherait à la mesure d'être prise, vous avez cité le cas de l'outre-mer, mais justement pour l'outre-mer, ce sont les présidents de collectivités qui émettront un avis cet avis, il peut être donné dans les heures qui suivent la constatation qu'il y a l'émergence d'un virus dangereux la symétrie ne peut pas être faite, elle pourrait l'être que je vous ferai une autre réponse, mais en l'occurrence ça se heurte à des difficultés pratiques réelles, alors je vous remercie de l'appréciation que vous avez bien voulu faire de notre travail, mais c'est justement en raison du caractère assez, je l'espère, approfondie du travail de la commission des lois que nous avons été obligés de vous faire cette réponse en étant navré de devoir vous la faire, mais si vous voulez retirer votre amendement, nous serons très heureux bien sûr. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, même avis madame la présidente, merci Monsieur K. Dick. Vous le retirez Monsieur K. Dick. Alors écoutez, moi je vous parlais juste d'un parallélisme des formes, d'accord, c'est que, avant de prendre une décision, c'est quelque chose que vous avez compris, pour les territoires d'outre-mer et là pour les Français de l'étranger, ça ne serait pas possible de les consulter avant, alors vous dites qu'il faudrait du temps pour réunir l'assemblée des Français à l'étranger, je vais vous faire un un aveu, une confidence, il existe de nos jours et c'est très utilisé la visio-conférence, et à l'Assemblée des Français, l'étranger, ils ont pris l'habitude, justement, de se réunir très vite, comme d'ailleurs les élus des Français de l'étranger et c'est comme ça que nous communiquions aujourd'hui entre nous, donc, pour répondre à votre juste et je trouve très pertinente remarque je veux vous faire passer un message qu'il y a un nouveau procédé aujourd'hui qui peut répondre à justement la vocation qui a été attribué au donc aux outre-mer, nous pouvons effectivement avoir cette réponse, c'est un principe républicain d'égalité qui se trouve juste entre la liberté, la fraternité et c'est ce que je réclame pour les Français de l'étranger, sinon ça donnerait l'impression que, il y a une France à part. Et ça c'est pas un principe républicain. Merci, merci. Alors donc je mets aux voix à Monsieur, le comte excusez-moi. Merci madame la présidente, le Sud-Ouest, mes chers collègues, sur le fond, j'ai la faiblesse de penser que notre mot l'amendement de notre collègue Chantrel qui proposait tout à l'heure, une consultation des conseillers des Français de l'étranger était plus adaptée, toutefois, monsieur le rapporteur, je me sens quand même très mal à l'aise avec votre réponse sommes-nous lorsque nous vivons à l'étranger des Français de catégorie B qui nous n'avons pas les mêmes droits, qui ne sommes pas digne d'être consultées lorsqu'on prend des décisions qui nous concernent. Eh bien non, en tout cas, nous revendiquons le fait d'être dans la communauté nationale à égalité et à partir de là, effectivement, il n'est pas illégitime qu'on nous pose des questions et on peut peut être aussi apporter des réponses et et à partir du moment où la pandémie est mondiale, ce n'est pas inutile de regarder au-delà des frontières. Monsieur le rapporteur. Non, madame la présidente, une consultation en visioconférence ne serait pas valable en l'occurrence, et il n'est pas précisée d'ailleurs dans cette tellement de monde que c'est ainsi qu'elle devrait être faite. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement de quinze qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

Madame le président, monsieur le ministre, chers collègues, je demande de remplacer le risque de saturation du système de santé par l'apparition de nouveaux variants constituant une menace sanitaire grave pour 2 raisons : dans le grand Hall de cet article concernant l'Hexagone on évoque l'apparition d'un possible variant de nouveau variant. Là c'est plus ça, c'est la saturation du système hospitalier, or cette structurelle, l'offre de soins chez nous et partout dans les outre-mer et structurellement insuffisante, c'est la raison pour laquelle je me suis opposé à l'amendement Mohamed et était au fil qui consiste à dire : vous êtes malade, vous ne pouvez même pas être soigné chez vous mais restez chez vous, c'est exactement le cas des Français résidant à l'étranger, restez chez vous, alors moi je demande une harmonisation pour éviter une inégalité de traitement, ce qui se fait ici dans l'Hexagone, c'est l'apparition d'un nouveau variant, je demande la même chose dans les outre-mer 2ème raison, c'est l'efficacité, pour être efficace, il faut aller vite, lorsque vous allez constater la possible saturation du système de santé, il sera trop tard, la pandémie sera là la circulation virale sera renforcée et bien présente et donc si on veut être efficace et de dire hé bien, pour l'égalité de traitement, éviter de faire des outre-mer des Français entièrement à part, il faut parler de nouveau variant. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Je regrette que ce soit celui des amendements de Monsieur Lurel qui arrive en premier, parce que la Commission a donné un avis favorable à tous les autres, j'y reviendrai tout à l'heure, mais pas à celui-ci, monsieur durer, j'en suis vraiment désolé, mais nous pensons effectivement que le bon critère pour restreindre l'accès à nos collectivités d'outre-mer, c'est le risque de saturation du système hospitalier pour une bonne et simple raison, c'est que lorsque ce risque survient, il est très grave, en métropole, si vous avez une saturation de l'hôpital de Mulhouse, vous pouvez faire des évacuations sanitaires à Strasbourg à Nancy à Metz ou dans d'autres villes, si vous avez dans votre collectivité une saturation de l'hôpital, vous ne pourrez pas faire d'évacuation sanitaire, donc c'est une mesure de sauvegarde et nous sommes là encore dans un cas très exceptionnels, je crois qu'il faut s'en tenir là, mais nous allons discuter d'autres amendements sur lesquels l'avis sera favorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur. Notre amendement vise à aligner les conditions du passe entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain sur celle du Pass entre le territoire national et l'étranger. Je suis favorable à ce que l'apparition et la circulation d'un nouveau variant soit également prise en compte sur l'instauration de ce dispositif lorsque cela s'avère nécessaire sur les déplacements entre territoires d'outre-mer, pardon les collectivités d'outre-mer, un territoire métropolitain, néanmoins je pense également que le critère de risque de saturation du système de santé quand même pertinent, c'est ce critère d'ailleurs sur lequel nous avons fondé les évacuations par pont aérien depuis la Polynésie, il y a quelques mois. En effet, le caractère insulaire des départements d'outre-mer rend les phénomènes de résurgence épidémique plus difficilement maîtrisable, s'ajoute à cela une offre de soins plus restreinte, c'est vrai, et une couverture vaccinale souvent moindres qu'en métropole, mais également des flux touristiques et des brassages de populations qui peuvent être très importants pendant l'été. Le critère de saturation du système de santé est alors nécessaire aux côtés de celui de l'apparition ou de la circulation d'un variant. Pour cette raison, je demande le retrait de votre amendement qui est en partie satisfait par l'adoption des amendements 55 et 65.

je ne veux pas évoquer des des situations personnelles lorsque on constatera que il y a saturation du système de santé, il sera trop tard. tard lorsqu'on l'a, on l'a déjà vécu, on a dû envoyer la réserve sanitaire, on a dû envoyer les armées mais le la circulation était bien là, en plus, c'est développer toute une propagande anti-vax, il était beaucoup trop tard, s'il faut attendre de constater ce qui existe en permanence l'insuffisance de l'offre de ce que la facturation presque permanente dans les hôpitaux des mer, il sera trop tard, je dis qu'il faut être efficace et aller vite et le constater le plus vite possible, voilà ce que je dis c'est pas plus compliqué que cela, on vient de faire quelque chose là, créé une sorte de prison sanitaire, vous ne pouvez pas être soigner chez vous, vous ne pouvez même pas ici en métropole je viens un peu cette situation particulière, je le dis très clairement condamné à à rester chez vous, vous n'avez pas de place, vous n'allez pas de soins, vous n'avez pas de médicaments, vous n'avez pas de soignants. Il sera un peu tard, moi je maintiens l'amendement parce que je connais un peu la la la, situation. Tu veux tout de même rassuré Monsieur Lurel on n'attend pas la saturation, c'est s'il y a un risque de saturation, les autorités sanitaires mettent en place ce filtrage, mais on n'attend pas la saturation, bien sûr, vous avez tout à fait raison Kant le le système hospitalier est saturé, il est déjà trop tard, mais quand on voit que les chiffres augmentent rapidement, on prend immédiatement la mesure. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 42 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui contrôle. Qui s'abstient n'est pas adopté un amendement 43 Monsieur Si madame la présidente, c'est un amendement simple hein, qui est de nature rédactionnelle pour intégrer toutes les natures d'exécutif de nos différentes collectivités dans les outre-mer. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Un avis favorable, madame la présidente. Si l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Monsieur le sénateur, je demande le retrait de votre amendement au profit de l'amendement quarante-cinq OK, je suis favorable et qui, dans sa rédaction prévoit les exécutifs locaux. Merci. Monsieur Lurel vous retirer non vous me demandez la parole ici. Non, madame la présidente, je ne retire pas les exécutifs locaux, j'ai 32 communes il y a à la tête de chaque commune un exécutif local, c'est le maire, j'ai eu un président de région, j'ai un président de département qui sont également des exécutifs locaux et donc, si on devait consulter tous les exécutifs locaux, on n'en sortira pas c'était pas efficace, je connais pas l'amendement que vous évoquiez, monsieur le Ministre, mais il me semble que cette rédaction est simple et on intègre la Guadeloupe qui a 2 exécutifs de collectivités dites majeures chez moi, régions et départements, c'est le cas de la Réunion mais ça peut être également en mettant le mot territoriaux, le cas de la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, c'est un autre sujet, ils sont autonomes en matière de, de, de santé, mais si vous mettez exécutifs locaux c'est vagues et c'est confus. Merci. Alors donc je mets aux voix l'amendement 43, qui a reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour, qui est contre qui. Abstient il est donc adopté l'amendement 58 hommes, madame la présidente Assassi. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, le dispositif choisi par le rapporteur dans le Sahara réécriture de l'article 2 circonscrit la possibilité pour le gouvernement d'exiger la présentation d'un certificat sanitaire de voyage pour les voyageurs ultramarins entrant sur le territoire métropolitain uniquement en cas de risque de saturation du système de santé en outre-mer s'il est prévu qu'en amont de toute implication du dispositif prévu l'exécutif de la collectivité concernés soient consultés, nous considérons pour notre part que ces derniers devraient être aussi pouvoir être à l'initiative de toute implication, je vous remercie. Merci la vue de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, chers collègues, nous avons inscrit à mon initiative, dans le texte de la commission des lois, un droit de propositions vous proposer un droit d'initiative, alors là, sans faire de juridisme, je suis obligé de vous dire que droit d'initiative des droits, de proposition, c'est pas exactement la même chose si on a votre amendement, on ne pourrait mettre en oeuvre la mesure qu'à l'initiative de la collectivité avec le droit de propositions, on permet à la collectivité, j'oserais dire de prendre l'initiative, c'est-à-dire de déclencher une décision mais qui ne lui appartient pas, qu'il appartient aux autorités sanitaires et je vous propose d'en rester au texte de la commission qui, à mon avis, ça satisfait très largement votre intention, vous n'avez sans doute pas entendu donner à la collectivité, le monopole de la démarche, donc si vous voulez bien retirer votre amendement vraiment la commission des lois vous en sera très reconnaissante. Merci monsieur le ministre avait du gouvernement même à vivre dans la presse, merci Monsieur Gay, vous le retirer. Merci beaucoup, l'amendement 45 a Monsieur Lurel. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, un collègue : c'est l'amendement présenté par notre collègue Concorde, bien entendu, accompagné par tout le groupe socialiste, écologiste et républicain, notre collègue propose au nom des exécutifs de donner cette décision à l'exécutif lui-même avec la précision qu'on vient d'adopter à l'exécutif lui-même et non plus. Par délibération. Puisque il faut au moins 12 jours pour convoquer une plénière alors qu'un président qui serait investi de pouvoirs propres pourrait faire cette demande-là et donc pour l'efficacité, là aussi, il faut aller vite, c'est ce que propose notre collègue Catherine Conconne et madame la présidente, si, si vous permettez, je présenterai aussi le hein, ça irait plus vite, elle propose que le 1er ministre répondent dans un délai de 10 jours pour que la chose soit pleinement efficace.

Favorable et sagesse, madame le président. Merci beaucoup. Alors je mets aux voix donc l'amendement quarante-cinq, qui a reçu un avis favorable de la commission et du gouvernement. C'est pour qui est contre. S'abstient et donc adopté et l'amendement 44 qui a reçu un avis favorable de la commission, avis de sagesse du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient donc adopté.

Je l'ai dit tout à l'heure, le résultat. Je vais juste signaler. Que sur l'article de chez une demande de scrutin public mais vous pouvez prendre la parole, je vous remercie. Tout à l'heure, je, je l'ai déjà signalé le le vote sur l'amendement consistant à ajouter le vaccin et le certificat de rétablissement était une des conditions du fait que nous puissions ou pas voter cet article 2, celui aussi sur les mineurs jusqu'à 18 ans, qui ne devait pas être soumis, on était une autre, ces 2 conditions n'ont pas été remplis, ce qui fait que nous ne voterons pas effectivement cet article de ce n'est pas la seule raison, il y en a une autre, c'est qu'en fait nous nous trouvons confrontés à une problématique qui reste toujours la même depuis que ces lois nous sort proposer c'est que sous couvert d'un besoin de réagir vite, un certain nombre de critères bien trop via trop floue de menace grave laissée à l'appréciation bien trop changeante du gouvernement et encore quand je dis du gouvernement, c'est pas de qui est-ce que c'est le comité scientifique, est ce que c'est le HAS est ce que c'est en fait le dernier qui a l'oreille de notre président, ce sont des éléments qui ne nous paraissent pas à des bases assez prévisible pour laisser l'exécutif décider seule de mesures si restrictive restrictive et pénalisante. Pour les mineurs, on l'a vu, qui ont déjà beaucoup souffert de la crise je j'aurais tendance à dire au gouvernement : occupez-vous plutôt de la qualité de l'air, des écoles, mais aussi, on l'a vu pour les Outre-Mer ou, ou, pour les Français de l'étranger, préparer l'urgence ne justifie pas tout, nous avons par le passé sur le sujet de la pandémie déjà légiféré en quelques jours et les mesures urgentes pour la restriction de liberté d'aller et venir existe déjà nous ne pensons pas nécessaire de donner trop de pouvoirs à l'exécutif, même si c'est pour un mois, avec retour de vol, Parlement, il suffit de regarder l'expérience avec l'avènement du variant brésilien ou le ministre des Transports de l'époque Monsieur Clément Beaune justifier du manque de concertation européenne pour m'attire les vols en provenance du Brésil, en assurant que le contrôle du motif impérieux et du PCR négatif suffisait suffit aussi de regarder l'argumentation de monsieur Véran face à l'anxiété des élus corses, la première été sur la demande de tests négatifs pas efficace, selon l'ancien ministre de la santé, comme l'a dit tout à l'heure de nos collègues, nous ne connaissons pas grand chose, mais nous voulons rester humble et donc nous ne voterons pas cet article de. Merci j'ai été saisi, comme je l'ai dit, d'une demande de scrutin public par le groupe, les républicains sur l'article de : il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Personne ne demande à voter, le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin numéro 120 sur l'article, le numéro de compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs, gros politique et notifié à la présidence Nombre de votants : 343 Nombre de suffrages exprimés 263 pour l'adoption 236 contre 27 Le Sénat a adopté. après l'article 2 je suis saisi d'un amendement le de rectifier de Monsieur mouillé. Merci madame la présidente, l'objet du présent amendement et de créer un comité national de concertation et de coordination des territoires pour la lutte contre le Covid 19, nous savons tous que durant la crise, les collectivités territoriales ont joué un rôle spécifique et ont montré une réactivité remarquables pour apporter une réponse adaptée aux besoins de concitoyens été l'amendement du sénateur Richard qui a été votée permet de créer une nouvelle autorité pour le suivi de la crise Covid Monsieur le Ministre, cet amendement est donc un amendement d'appel pour que les associations représentant des collectivités, les parlementaires soient associés à cette nouvelle instance, je porte ici une demande forte des collectivités et notamment de l'Assemblée des départements de France, je vous remercie. C'est une demande de retrait, chers collègues, bien que je comprenne parfaitement le l'intention mais si vous voulez qu'on passe au vote, je m'en remettrai à la sagesse, mais il nous semble que il y a déjà de multiples consultations possible qu'elles sont d'ailleurs nécessaire, qui n'est pas indispensable d'en ajouter d'autres, sachez que la commission des lois, est extrêmement sensible à la nécessité de prendre en compte l'avis des élus qui savent la réalité de la situation dans leur collectivité. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, votre amendement vise à proposer la création d'un comité national placé auprès de la Première ministre pour associer les collectivités à la lutte contre le Covid 19. Je partage votre souci d'associer les collectivités territoriales, aux prises de décision en temps de crise sanitaire, même si les décisions à prendre un pause d'agir avec rapidité et efficacité, à la fois au niveau national, mais également dans chaque territoire autour du préfet et du directeur général de l'Agence Régionale de Santé les élus et acteurs de terrain ont été associés. Mais le comité que vous appelez de vos voeux existe déjà sous une forme très voisine avec le comité de liaison et de contrôle instituer à l'article 11 de la loi du 11 mars 2020 que le présent projet de loi maintient dans tous ces éléments pour cette raison, votre amendement me semble satisfait. Merci monsieur mouillé, il faut le retirer. Oui, oui, bien sûr, je retire parce que j'ai évoqué que c'était un moment d'appel simplement Monsieur le Ministre, j'entends votre argument et cet amendement a été rédigé avant la la possibilité d'installer une nouvelle instance de suivi et donc ma caution c'est quel sera le lien entre ces instances scientifiques et les collectivités voilà donc j'aurais souhaité une réponse de la part Monsieur le Ministre, ce lien particulier je retire l'amendement bien sûr.

Merci madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, monsieur le ministre, hier, l'Académie de médecine à donner son avis sur la réintégration des soignants non vaccinés, avançant un risque de perte de cohésion et de confiance entre malades et soignants, il me semble inapproprié de parler de confiance alors que des feux font rage dans plusieurs régions de France, que des femmes et des hommes sont poignardé en pleine rue, nous continuons d'exclure des professionnels investi pour la sécurité de leurs concitoyens, alors que l'hôpital est la queue ni nous continuons d'exclure des soignants alors que, alors même que. Nous avons été autorisé des personnels malades mais à exercer auprès des patients, il a été reconnu que le vaccin n'empêche pas la contamination et la vague que nous avons connu après la mise en place du Pass vaccinal le démontre aujourd'hui ce projet de loi lève le passe vaccinal sur le territoire hexagonal et c'est enfin monsieur le rapporteur, un souffle de liberté mais c'est surtout la fin d'un dispositif injuste, inéquitable et parfaitement contreproductif cet article 2 bis, a pour objet de rétablir un peu de cohérence en permettant aux agents publics non vaccinés de réintégrer leur emploi dans des modalités qui ne constitue pas une charge supplémentaire pour l'État, il en va de la santé et de la sécurité des Français, il en va de la cohérence scientifique, mes chers collègues, pour protéger l'hôpital nous avons fermé des Français aujourd'hui pour protéger les Français, nous, nous, nous, nous, nous vous demandons, monsieur le Ministre de libérer nos soignants nos forces de l'ordre nos pompiers 140 professionnels et 5000 volontaires et nous en avons besoin.

bon ce de bis introduit un principe de réintégration des personnels suspendu, j'aimerais pouvoir dire et redire devant vous ce soir que je crois à la science à la médecine et au progrès les bon de le répéter, je suis pour la vaccination car elle sauve des vies, c'est mon seul souci, il me plaît de vous dire et de vous redire que je ne suis pas opposé à la réintégration des personnels suspendu comment refuser un agent hospitalier suspendu d'être réintégré par exemple dans les jardins d'un hôpital. Je me vois mal aller Dieu c'est pas possible, bien, je reste opposé à la réintégration des personnels suspendu des soignants non vaccinés au chevet des malades. Ou des personnes fragiles ou vulnérables. J'affirme ici de manière, comme dirait Césaire autre lucide et conséquente. Que je reste opposé à cette réintégration. Je reste opposé, c'est une exigence morale. Celle de l'exemplarité et de l'éthique attaché aux soins et je rappellerai et je n'aurais pas le répéter dans la présentation de l'argument si j'ai encore quelques minutes au niveau national, il y a 500 infirmiers qui serait suspendu pour 263000 infirmiers 75 médecins et pharmaciens pour 85000 médecins 200 pompiers sur 40000 vous avez eu IV avis puisque le ministre nous dit : je veux un avis éclairé pour objectiver la situation elle est déjà objectiver puisque vous avez l'avis du comité scientifique fermement opposé, la vie de l'Académie de médecine, la Fédération hospitalière de France, le Conseil national de l'Ordre des infirmiers, je finis Madame le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers voilà. Merci. La parole est à monsieur Georges Patient. La vaccination est encore plus obligation vaccinale pour les personnels de santé ont été très mal accueillis en Guyane pour ne pas dire plus, je crois pouvoir dire qu'il en a été de même dans d'autre côté risquera ultramarins l'obligation vaccinale en dépit des des virulente contestation a finalement été appliqué avec les sanctions prévues en cas de non-vaccination au dernier décompte en Guyane, il y avait craint quatre-vingt-six personnes suspendue pour non-vaccination, les taux de vaccination, ils sont toujours à des niveaux encore insatisfaisant, entre 75 et 88 % aussi l'état des connaissances progressant tout comme la prise en charge des malades, il convient dès lors de réévaluer la pertinence de l'obligation vaccinale, si l'on estime que le risque n'existe plus, ou du moins qu'il est faible, alors il faudra suspendre la mesure, c'est ce que propose cet article additionnel, mais c'est également ce que, sans vouloir faire le gouvernement puisqu'il a saisi sur ce sujet, la Haute autorité de santé la semaine dernière. cas d'avis négatifs de la côte, autorité de santé, il faudra néanmoins donner des perspectives à ces personnels, quitte à imaginer imaginer des mêmes aménagement de leur activité, nous ne pouvons la laisser indéfiniment sans travail pouvoir nous même nous le permettre, à l'heure où nombre de nos services d'urgence sont en souffrance, au moment où je vous parle, je pense notamment au centre hospitalier de l'ouest guyanais qui ne fonctionne pas la nuit, faute de personnel suffisant, je vous en remercie. Merci madame Sylviane Noël merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Comme vous le savez, je me bats depuis maintenant un an quasiment en faveur de l'abrogation de l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers, et je suis heureuse que ce sujet prenne enfin toute sa passe dans le débat public, enfin, car cette mesure en oeuvre depuis presque un an, a fortement déstabilisé notre système de soins et de secours face à certains qui tentent de minimiser les chiffres, évoquant que les soignants suspendus ne représenteraient que 0,53 % de nos effectifs de santé que les pompiers suspendus ne représenteraient que 2 % des effectifs il combien une bonne fois pour toutes de rétablir la vérité sur ces chiffres très fortement sous-estimé qu'ils ne prennent pas en compte tous les soignants qui ont démissionné de la fonction publique, tous ceux qui ont demandé une mise en disponibilité, tous les professionnels libéraux, les médecins généralistes, les sages-femmes, les kinés qui ne relèvent pas de la fonction publique hospitalière et qui ne sont donc pas suspendu, ils sont interdits d'exercice, monsieur le Ministre donnez-nous des chiffres de vrais chiffres alors que notre hôpital est à l'agonie, alors que la France brûle, au sens propre comme au sens figuré, nous nous payons le luxe aujourd'hui de nous passer de milliers de soignants et de pompiers qui ont juste voulu exercer leur libre choix, comme n'importe quel Français à l'égard d'un vaccin qui ne protège ni de la contamination, ni de la transmission du virus, il n'y a plus rien de sanitaire, ni de scientifiques dans tout cela, nous sommes face à une obstination aveugle dogmatique et idéologique qui nous conduit dans le mur, monsieur le rapporteur, dans ces conditions, permettez moi de juger, même si je me réjouis de votre amendement que votre amendement traitant de ce sujet est beaucoup trop timide vous laisser une nouvelle fois la main au gouvernement pour procéder à cette réintégration lorsque les conditions seront réunies, pardon, mais c'est à nous, députés et sénateurs de le faire et de le décider maintenant cette obligation vaccinale, elle a été mise en oeuvre par la loi, ce qu'une loi peut faire une loi peut le défaire, il ne faut pas perdre une minute, la situation est trop grave et ce sera donc le sens d'un de mes amendements. Merci monsieur le questeur Jean-Pierre Sueur. je dois remercier Marie-Noëlle Lienemann qui tout à l'heure a dit avec tellement de force, ce que les vaccins apporter à la science, la médecine et la vie tout simplement, de dizaines et centaines de millions de personnes, je crois que c'est très important de le redire je voulais intervenir simplement sur une question qui paraîtra formelle, mais je me souviens du jour funeste où la conférence des présidents du Sénat a décidé que tous les rapporteurs seraient désormais tenus dans l'exercice de leur mission de déclarer devant la commission un périmètre au sein duquel on aurait le droit de déposer des amendements et à l'extérieur duquel les cependant seraient bannis, j'ai toujours été contre cette procédure qui est attentatoire aux droits du Parlement qui me paraît d'ailleurs poser un problème constitutionnel, eu égard au droit mais je sais qu'il existe, l'article 45 et sans doute a-t-on voulu prévenir les décisions éventuelles du Conseil constitutionnel, qui est très, très rude sur cette question et alors je me suis étonné : je m'étonne aussi en séance publique, que cet article 2 bis, il est le fruit d'un amendement. Soit apparue. Alors que le texte tel qu'il nous a été présenté. Ne permet pas de traiter de cette question, c'est autre chose, alors, naturellement, j'ai entendu la réponse de monsieur le rapporteur, je sais qu'il la rappelle rappellera ici, je le suppose, mais je vous assure que cet épisode montre tout simplement le caractère très arbitraire dans lequel on peut tomber avec ce type de procédure. Merci monsieur Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, chers collègues, tous les articles sont importants, cet article, simplement je souhaitais intervenir modestement concernant cet article 2 2 bis qui fait référence à la loi du 5 août 2000 21 ans, n'oublions pas de rappeler bah tout le travail qui a fait la commission des lois depuis mars 2020 dès le premier confinement, il y a eu aussi beaucoup, beaucoup particulièrement sensibles dramatique et cette loi qui fait référence à la gestion de la crise sanitaire, loi du 5 août 2021, certes il y a des amendements et je crois que toutes tous les amendements sont toujours à la fois intéressants et qui suscite aussi des débats, des réactions et je crois que mérite aussi du respect, il y a certes des amendements concernant cet article 2 bis de suppression, il y a aussi et surtout des amendements qui visent à réintégrer les agents en fonction publique ou autre bien entendu les personnels soignants, suspendu, en effet, des milliers de soignants, les sapeurs-pompiers, forces de sécurité qui sont concernés et qui ont été aussi depuis plus de 2 ans, particulièrement très sollicité beaucoup de collègues ont rappelé aussi les besoins en personnel, au niveau des des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, tous les établissements de de soins de santé, et c'est vrai que les sapeurs-pompiers qui sont aussi et toutes les forces de sécurité très, très sollicité encore plus en ce moment on est mérite aussi bien entendu notre respect de notre reconnaissance, sujet hautement sensible mais d'un souci je dirais de essayer de trouver le bon sens et c'est vraiment très, très compliqué, donc je j'écouterai avec attention les avis du rapporteur de la commission des lois pour me pour le vote concernant cet article 2 bis merci beaucoup. Merci Madame Cécile Cukierman. nombreux, ici, qui ont toujours été convaincus que le vaccin à défaut de solder cette pandémie était en tout cas une arme efficace pour empêcher sa propagation, et notamment le développement des formes les plus graves qui ont amené malheureusement un certain nombre de nos compatriotes soient à soit à souffrir encore aujourd'hui de des séquelles et y compris du Covid long qui n'est toujours pas reconnu cependant sur la question des personnels tant de santé que des sapeurs pompiers, nous mesurons maintenant le le temps faisant la difficulté qui peut d'abord faire preuve d'une incompréhension. Le Pass vaccinal n'existe plus, il y a donc aujourd'hui des sapeurs-pompiers qui sont vaccinés qui sont en possession d'un schéma vaccinal complet qui pour autant sont porteurs du virus, nous avons des personnels qui sont

donc je crois que nous avons réellement à réfléchir, et la question n'est pas là dans une vision jusqu'au-boutiste mais nous avons besoin en métropole comme dans les outre-mer, de ces femmes et de ces hommes de personnel soignant de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires pour répondre aux urgences de cet été, moi je ne souhaite pas que ce soit le gouvernement qui décide, je pense, ça va être autre Parlement justement de décider comment les réintégrer, avec des tests avant la prise de service sur certains postes de service, plutôt que d'autres mais en tout état de cause, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur ne pouvons soutenir cet article. Telle que rédigée merci monsieur Alain Milon. Merci madame la présidente, je voulais intervenir parce que je ne voterai pas cet article 2 bis et je voterai évidemment les amendements de suppression qui seront présentées par mes collègues, je voudrais dire simplement plusieurs choses en voyant cet article j'ai emmené discuter discuté avec le rapporteur, hier encore, je me suis interrogé sur le personnel médical et sur le personnel médical non vaccinés, j'ai repris les chiffres de la région Provence Côte d'Azur

médecins et personnel médical de ces sanitaire de ces hôpitaux et sur l'ensemble des personnels soignants des maisons de retraite, nous avons en tout et pour tout, sur la région PACA exactement selon l'ARS, 264 personnel suspendus sur les milliers de personnes qui travaillent dans les hôpitaux et dans les hospices, c'est c'est vraiment des gens qui refusent la vaccination et les et les réintroduire ces réintroduire des gens qui refusent la vaccination et c'est donc permettre de faire un précédent avec des gens qui, lorsqu'ils seront pourraient être embauchée à l'hôpital doivent être vaccinés contre l'hépatite doivent être vaccinés comptait Thanos refuseront ce genre de vaccination et si on leur refuse l'entrée dans l'hôpital parce qu'il refuse de tétanos, c'est l'hépatite, ils iront vers un juge et le juge pourra s'appuyer sur le précédent que vous créez aujourd'hui donc, vraiment, comme l'a dit Madame Guillotin dans son intervention, il y a un risque majeur de créer une je une je sais pas si le terme exact, mais une jurisprudence en tout cas un précédent extrêmement important et comment allez-vous faire après pour les parents qui refusent la vaccination pour leurs enfants sur la rougeole pour les refuser en crèche ou à l'école, comment allez-vous faire pour les parents qui refusent le papilloma virus la vaccination contre le palu m'avait papilloma virus, nous créons un précédent extrêmement dangereux, je voterai contre l'article 2 bis et évidemment les amendements de suppression. Merci, cher collègue Madame Raymonde Poncet Monge. Merci madame la présidente, alors moi aussi, en préalable, hein, je rappelle que la crise Covid a poussé le gouvernement à lancer une vaste campagne de vaccination largement suivie et qui a permis de sauver de nombreuses vies bien la vaccination a été rendue obligatoire pour les soignants et les sapeurs pompiers, mais nous avons à juste titre ici refusé le licenciement des personnes qui, alors en poste, hein, c'est pas à l'embauche, alors en poste, refusaient la vaccination créant dès lors un OFNI législative dans le droit du travail, une suspension sans rémunération pour un motif nouveau interdisant le licenciement n'obligeant pas la démission, on estimait, vous l'avez dit est-ce l'an passé à 15000 le nombre des soignants concernés 2 tiers auraient été réintégré bien mais que faire de ce qui reste ces soignants vont-ils rester suspendu ad vitam eternam, sans vision sur les conditions de leur réintégration à part la vaccination, bien sûr, il faut donc éclaircir les critères qui justifie de maintenir cette suspension en fait les mêmes, qui est du maintien de l'obligation puisque nous savons que nous allons désormais vivre avec la Covid, les raisons qui nous ont fait adopter l'article hein, ah, nous conduisent à poser légitimement cette question quand, faute de soignants quand même des soignants vaccinés mais contaminés sont autorisés à exercer voir sont rappelés, je suppose qu'on a examiné le calcul bénéfice risque qu'on juge alors suffisantes les mesures barrières, il est temps de réinterroger c'est légitime la suspension, encore en vigueur de centaines d'infirmiers est-ce toujours impératif et justifiée en regard des risques nosocomiale et sur quels critères ont jugé nous devons trancher à moins de vouloir punir à avis des soignants qui ont refusé une sorte de bannissement, j'entends cela un petit peu chez certains décidé alors dans ce cas-là, il fallait les licenciés, il faut être cohérent des et décidé sur

Merci madame la présidente, alors je voudrais à ce stade, attirer l'attention sur les personnels qui sont vaccinés, parce que ce sont des personnes qui met aussi en danger parce qu'ils sont pour la plupart en burn-out ça ce sont des personnes fatiguées, épuisées, pour la plupart, donc je pense qu'il faut aussi humaniser notre démarche, ce sont des personnes qui sont en souffrance et qui ne peuvent pas prendre leurs congés leur récupération, voilà tout simplement ce que je voulais dire. Merci, Oui, chers collègues, j'entends certains collègues s'émouvoir des démissions de l'hôpital public, on aurait été terrassé brutalement l'hôpital n'aurait pu le personnel à cause des refus de vaccination, j'aurais aimé, chers collègues, que vous soyez plus mobilisés Kant avec mon groupe et beaucoup d'autres, nous demandions à l'état de recruter dans les hôpitaux de mieux rémunérer les soignants et les personnels et d'avoir un plan si je puis dire, Marshall pour être rapide pour sauver les hôpitaux là on vous entendait pas, c'était pas grave si on pouvait s'arranger, mais maintenant, il y aurait tous les maux de l'hôpitaux des hôpitaux viendrait de du fait qu'il y a pas de soignants es trop de soignants qui ont refusé la la vaccination,

entre le libre arbitre de chacun la responsabilité qu'il prend pour l'assumer et la loi générale qui s'impose à tous, hé ben nous savons de beaucoup de soucis à nous faire parce que c'est la crise de l'intérêt général qui s'exprime à partir du moment où nous avons décidé, pour des raisons de protection, et quand on est malade soi même, on est quand même plutôt rassuré de penser que les personnels sont vaccinés, même si lucidement, on sait que c'est pas à 0 risque, c'est le principe dit de précaution. Il faut prendre toutes les précautions possibles, même si elles ne sont pas absolues, donc moi je crois que si on commence à mettre le doigt dans l'engrenage que chacun décide que c'est bien fondé ou pas, on peut contester la loi moi je comprends certains la conteste parce qu'ils sont pas d'accord, il dit : ça sert à rien, mais, mais moi je crois que nous avons intérêt à défendre pied à pied les principes que nous avons défait la fonction publique, c'est des responsabilité qu'on assume des contraintes de liberté et un certain nombre de d'Avantage du statut tout moi je, je vous demande de ne pas accepter la réintégration des soignants.

de ce que représente l'effectif réel fonction publique hospitalière salariés de droit privé, profession volons pompiers professionnels et volontaires pour qu'on sache vraiment dans le pays à l'instant où on se parle, vous devez les éléments statistiques qui vous permettent de répondre à cette question Monsieur le Ministre, mais de ne jamais

2ème chose je remercie le rapporteur puisque avec son amendement, il permet, et qu'on est que ce débat ait lieu. Parce que que je sache, je n'ai pas mémoire nous ayons décidé ici pour ceux qui l'ont voté pour, ceux qui ont voté la suspension des soignants non vaccinés que nous les ayons suspendu a dit Amsterdam et Antoine Flahault, professeur de médecine à Genève, dit le maintien de la suspension des soignants non vaccinés n'est plus fondée sur surveillance autres plan scientifique il y a, en effet, il n'y a en effet pas de raison d'exiger le vaccin chez les soignants, car il n'évite pas ni ne réduit pas suffisamment les contaminations des nouveaux variants du Sars CoV 2 sur un plan éthique, il n'y a pas davantage de raisons de ne pas réintégrer les personnes non vaccinées parce qu'il pense très différemment des vaccinés mais c'est une condition de leur embauche que d'avoir des raisonnements scientifiques validées par le gouvernement ne pas réintégrer les non vaccinés sans un minimum de de fondement scientifique créerait un précédent questionnable en termes de gestion des fonctionnaires blâmer ses personnels de santé. Je cite toujours pour leur comportement passé irresponsable et illégal, oui c'est Flo qui parle, ne pas les réintégrer non Antoine Flahault, professeur de médecine, personne qui a eu énormément intervenu pendant le débat si cher collègue. Donc, 2 amendements que nous allons étudier identique et faisant l'objet d'une discussion commune donc, et ce sont des amendements de suppression et le 1er 52 madame dit autant. Merci madame la présidente, à nouveau, je crois que tout a tout a été dit pour expliquer le la suppression de de cet amendement et qui qui remet en cause le principe de réintégration des des soignants non vaccinés déjà c'est une modification du du régime d'obligation vaccinale qui a été décidé à un moment où la crise sanitaire été là, on parle bien d'obligation vaccinale et la situation sanitaire aujourd'hui, on l'a dit tous dans cet hémicycle n'est pas derrière nous, mais encore en situation d'épidémie et cette obligation vaccinale des soignants ma perdure, et je crois que la moindre des choses pour un soignant, c'est de la respecter, je crois, comme certains l'ont dit à la foi en la science, bien évidemment, la médecine, mais surtout en l'intérêt général et je ne pense pas que chacun, dans une société dans un métier dans un établissement puisse décider

plusieurs ici l'ont fait, moi si j'avais pas mon certificat de vaccination contre l'hépatite B, enfin je pense que tout le monde était pareil hé ben, nous ne faisions pas de stage, c'est-à-dire je ne rentrez pas en médecine ont demandé, donc c'est rien n'a changé en fait dans le système, on a un débat aujourd'hui sur cette réintégration, alors qu'il un débat sur le fait : est-ce qu'aujourd'hui la vaccination des soignants est encore nécessaire, ça c'est un débat qu'il faudra voir si elle n'est pas nécessaire, hé ben on a on annule cette cette obligation vaccinale, hé bien évidemment que les soignants non vaccinés sont réintégrés, mais si la science, la médecine, enfin les les autorités sanitaires et Monsieur le Ministre, va peut-être nous nous informer des contacts qu'il a eu, mais si cette juste cette vaccination, vu le contexte sanitaire est encore obligatoire, les soignants non vaccinés ne peuvent pas être en contact avec des patients, notamment les plus fragiles dans des services de réa où on sait que 9 patients sur 10 sont des patients non vaccinés, donc je j'en dirais pas beaucoup plus, tout, tout a été dit, je vous remercie, Madame Lienemann, d'ailleurs, pour le petit coup de gueule que vous avez eu tout à l'heure parce que juste 2 choses, c'est pas en répétant des choses fausses sans cesse qu'elle devienne vrai. Merci l'amendement soixante Madame Cohen. Oui merci madame la présidente, mes chers collègues, avec cet article 2 bis. Le rapporteur propose une issue à la situation des personnels soignants, suspendus en leur permettant en fait d'être réintégré dès lors que la situation épidémique épidémiologique constaté par la Haute autorité de santé ne nécessiterait plus l'obligation vaccinale pour ses personnels, je veux saluer cet effort de réécriture de la part du rapporteur Philippe Bas, il s'agit effectivement d'une légère avancée par rapport au texte initial du gouvernement mais il nous paraît difficile au niveau de notre groupe majoritairement de laisser les personnels de santé, suspendu à cette évolution qui semble s'inscrire sur le long terme et moi je pense que le débat là devient plus intéressant parce qu'il est moins binaire, je pense que, en tout cas je fais partie de ceux des ceux qui, trouvant que la vaccination, c'est une arme efficace pour combattre effectivement cette pandémie, même si ça a été dit c'est pas suffisant, mais en tout cas c'est une manière de protéger les personnes, les patientes et les patients, mais on sait également les limites au niveau de la contamination et puis là, quand on parle des personnels merci, mes chers collègues, on s'attaque quand même au droit du travail et ça c'est une première, si je puis dire, c'est-à-dire que est-ce que ces personnels qui sont des, des, des personnels de santé, qui sont des pompiers est-ce que finalement ils vont être intégrés ou c'est ils sont suspendus ad vitam eternam, enfin c'est pas possible, et en même temps on nous dit : oui mais c'est important : ils doivent prendre leurs responsabilités, mais est-ce que vis-à-vis de toutes les responsabilités sont prises quand on demande au personnel soignant, alors qu'ils ont le Covid d'aller travailler, parce qu'il manque du personnel, là on ne s'occupe pas des problèmes de contamination, là on ne s'occupe pas de leur santé, donc on peut pas faire 2 poids 2 mesures et il me semble important de dire aujourd'hui que, y compris continue de la situation de nos hôpitaux des établissements publics de santé il est important de réintégrer ces personnels, je vous remercie. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, c'est pas grave. Madame la présidente, les amendements dont il est question ici. Porte sur la suppression d'une disposition adoptée. Par la commission des lois qui ne prévoit pas la réintégration. Des personnes non vaccinées. Je tiens à le dire parce que la plupart des interventions qui ont eu lieu. étaient soit contre la réintégration soit pour la réintégration. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, vous pouvez d'ailleurs renouveler votre prise de position dans un instant parce qu'il y a bien des amendements. Qui exige, selon des modalités différentes, d'ailleurs la réintégration. Je n'ai pas proposé la réintégration à la commission des lois, la commission des lois n'a pas adopté d'amendements. Procédant à la réintégration. Le Sénat a voté l'obligation vaccinale. Le Sénat a également voté la suspension d'activité des personnels soignants principalement qui n'étaient pas vaccinées dans le but de protéger les malades. Les personnes âgées, les personnes handicapées en établissement médico-social, je tiens à ce que les choses soient claires. Parce que c'est ainsi qu'elle se présente. Mais à la différence des vaccinations qui sont nécessaires pour l'accès à la fonction publique hospitalière, la vaccination contre le Covid est une vaccination temporaire, les personnels qui n'ont pas voulu se faire vacciner n'ont pas été licencié. Leurs Liens avec le service public hospitalier ou avec une clinique ou un établissement médico-social privé n'est pas rompu. La suspension du contrat de travail est par définition temporaire et non définitive. Que tous nos collègues qui pensent qu'on pourrait ne jamais réintégrer ses personnels le savent bien. Le droit applicable avant la proposition adoptée par la commission des lois. Exclu. Qu'il reste suspendu pendant toute la vie si on avait voulu les écarter définitivement de leur métier pour des raisons qui tiennent à une sorte de morale cas personnel soignant ne devrait pas refuser de se faire vacciner parce qu'il expose des patients à un risque que tous ses collègues sachent bien que cette exigence morale tout à fait respectable qu'il voudrait voir imposer n'est pas dans le droit positif actuellement applicable. Donc, tous ont vocation à reprendre un jour leur travail est ce que nous proposons, où ne devons proposer qu'ils reprennent maintenant. Je réponds : non. Est ce que nous devons prévoir les conditions dans lesquelles ils le reprendront je réponds oui, et c'est d'ailleurs ce que la commission des lois fait. Parce qu'actuellement c'est un pouvoir discrétionnaire du gouvernement ne pouvons faire confiance au gouvernement ou ne pas lui faire confiance, en tout cas sa liberté d'action est totale. Et nous avons pensé, face à un sujet qui effectivement ne concerne pas de nombreux agents. Mais un peu plus de 2000, c'est-à-dire très peu d'agents à l'échelle de l'emploi de plus d'un 1000000 de personnes au sein du service public hospitalier et des cliniques privées. Hé bien, ces quelques centaines de personnes, elles ont droit à des égards : elles ont droit à ce qu'on s'occupe d'elle. On n'a pas voulu qu'elle contamine la cause est entendue : mais enfin, elles ont une vie, une famille à revenus à acquérir par leur travail, il est bon d'organiser leur retour et de ne pas laisser ce retour à la discrétion du gouvernement : nous voulons que une décision médicale s'impose au gouvernement. c'est la seule chose que nous ayons décidé alors nous avons dit, je pense que c'est pertinent que c'est la Haute autorité de santé qui prendra la décision de dire ça y est enfin libre. Le Covid c'est fini l'obligation vite vaccinal n'a plus de sens pour le Covid et puis ce qu'elle n'a plus de sens, le lendemain, Monsieur le ministre. Vous serez en tort, si vous ne prenez pas le décret autorisant la réintégration et pour être sûr que cette haute autorité de santé. Se prononce. Au moment opportun et que les choses ne traînent pas dans la situation, ce sera absolument améliorer, nous disons que la Haute autorité peut s'autosaisir, que le gouvernement peut la saisir que le nouveau conseil qui se substituera au conseil scientifique peut la saisir, mais aussi que les commissions des affaires sociales de nos deux assemblées auquel je crois Monsieur Alain Millon qui s'est exprimé tout à l'heure peut faire confiance, comme nous tous pourront saisir la Haute autorité de santé, c'est tout, rien de plus et rien de moins, et c'est déjà un pas en avant pour dire assez personnels, moi je pense qu'ils ont eu tort de ne pas se faire vacciner mais ils avaient la liberté de ne pas se faire vacciner, car on ne vaccine pas de force en France. En revanche, nous avons voulu mettre à l'abri les malades, les personnes âgées, les personnes handicapées et donc ils n'ont pas pu rester au contact de ceux-ci, pas plus que les pompiers qui actionnent les secours d'urgence, et par conséquent nous sommes maintenant, je crois, dans une situation, je le dis très sobrement, où il y a un chemin vers la réintégration de ces centaines d'agents qui n'ont pas reçu une punition mais qui se sont vu imposer de ne pas faire prendre de risques aux malades et aux personnes vulnérables, il y a un chemin, nous le créons mais nous ne créons pas de manière fantaisiste en disant scrogneugneu je décide aujourd'hui, moi, sénateur de les réintégrer parce que ceux-ci n'a pas de sens, je crois que la décision doit être médical, elle le sera, et c'est la raison pour laquelle je vous demande de rejeter la suppression de notre article 2 bis et puis tout à l'heure, je voudrais demanderait également de rejeter la réintégration, c'est le souci d'équilibre et de mesures dont on a une certaine pratique au Sénat. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est minuit passé. Alors je vous propose de prolonger notre séance afin d'achever l'examen de ce texte. Je ne vois pas d'observation, il en est ainsi décidé. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, la commission des lois a retenu un dispositif équilibré sur les conditions d'une levée le moment venu de l'obligation vaccinale facilitant notamment la saisine de la Haute autorité de santé pour se prononcer sur son bien fondé, je vous ai parlé tout à l'heure de transparence, je vais donc être transparent sur les derniers chiffres en ma possession concernant le secteur sanitaire. de personnels soignants et non soignants parmi ces suspensions 75 médecins 32 sage-femme 608 infirmière 600 une aide-soignante et 52 kiné. La ville du gouvernement est donc défavorable à la suppression de cet article, introduit par la commission des lois. Merci. Alors avant de donner la parole pour explication de vote, je voulais juste informé l'assemblée que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains je donne la parole à Monsieur Théophile. La la ministre et chers collègues, je ne voulais pas intervenir sur ce sujet puisque ce sujet a fait de gros dégâts, de très gros dégâts chez nous et qui continue, je suis de la Guadeloupe. Je sais que 94 à 95 % des soignants sont vaccinés, chez nous il reste Delta mais je vais donnant Ratio ratio de taux de chômage, il y a à peu près 180. Personne à 200 personnes qui sont devant le CHU. Et qui ont décidé de d'enfer domicile depuis quelques mois, c'est toute la Guadeloupe à peu près qui passe le matin devant le CHU pour soit donné à manger soit laissé quelques dit euros pour que ces personnes puissent en tout car s'occuper de leurs enfants pendant la période électorale et vous savez, chez nous 200 personnes ça touche rapidement toute la Guadeloupe, ils ont décidé les Guadeloupéens de faire la peau, de tout ce qui ne sous ne tenait pas hé bien les suspendu, faire la faire la peau politique, c'est devenu un sujet national tout ceux qui était et qui prônait la la non réintégration des soignants ont été battus et ça, c'est un pan 2ème chose je parlais du taux de chômage, hé bien ces personne n'a ne travaille pas et n'ont pas de revenus et c'est ce qui rythme la vie aujourd'hui en Guadeloupe, ce que je demande, pourtant je suis un défenseur du vaccin, j'en ai trois et très rapidement. J'étais président de la Fédération hospitalière des Antilles et de la Guyane, je connais, comment ça se passe, je suis je suis rationnel. Ce que je demande c'est qu'il y ait, et c'est une proposition,

parce que tant que l'épidémie continuera et des vagues sont à venir, hé bien l'obligation vaccinale des soignants sera maintenu et cet cet article 2 bis ne propose pas de réintégrer des personnes alors que l'obligation vaccinale est en vigueur, il faut être cohérent, si on veut que ces soignants reprennent leur travail, il faut soit levé l'obligation vaccinale et je n'ai pas entendu qu'il en soit, question. Soit, sinon abattre. Abattre une valeur fondamentale de l'engagement dans un métier de soignant, qui est d'accepter de se plier à des règles de protection collective de solidarité réciproque au-delà de son propre choix individuels, et si cette porte est ouverte, hé bien les dégâts seront considérables dans notre société. Confronté à cette question. Il eut été plus sage de s'en tenir au dispositif actuel qui prévoit que par décret après avis de la Haute autorité de santé l'obligation vaccinale puisse être levées et donc logiquement les gens être intégré mais le rapporteur a choisi d'étendre le Champ du projet de loi et on verra bien, éventuellement ce que le conseil constitutionnel en dira pour traiter cette question. ça n'apporte rien de plus, ce n'est qu'un message politique qui est envoyé et qui prend place et Patrick Kanner, l'a dit, dans le cadre des nouveaux équilibres politiques de nos assemblées et nous avons même assisté aujourd'hui dans notre hémicycle à un retrait par le groupe, qui soutient toujours le gouvernement d'un amendement contre l'avis du gouvernement, mais pour faire passer le texte avec la majorité LR du Sénat, pourquoi pas, mais il faut le dire clairement, ce n'est pas une posture scientifique ou autre, c'est un choix politique. Merci Monsieur Chassaing. Donc je dans le sens de ce que vient de dire Bernard Jomier, si vous voulez la la réintégration du personnel ne peut pas être enfin tout de suite d'ailleurs, elle sera faite par la par si l'évolution de la situation épidémiologique le justifie donc c'est pas du tout pour pour l'instant, mais en fait je voterai l'amendement de Madame Guillotin Véronique Guillotin, pourquoi, parce que si vous voulez, on retrouve, on retrouve à l'article 12 de la loi du 5 août 2021, le point cap qui permet au gouvernement par décret après avis de la chaise de réintégrer tout ou partie des soignants non vaccinés après avoir voté l'article 2 bis, ça pourrait être fait par la chaise seul mais déjà, ça peut être fait dans le cadre de la loi du 5 août 2021.

Madame Müller Bronn oui, merci, madame la présidente, je ne. C'est pas très longue, mais concernant le le personnel soignant dans ce ce mot qui englobe soignants et il y a des personnels administratifs, on a tous rencontré des personnels administratifs des hôpitaux, des centres médico-sociaux qui sont aussi touchés par l'interdiction d'exercer, or ils ne sont pas en contact avec les malades, moi je, on a reçu par exemple des des pédopsychiatres qui travaille avec les établissements scolaires qui prennent les enfants dans une salle de 20 mètres carré et qui sont à distance d'un enfant, alors que cet enfant va être avec 30 autres enfants dans une salle de classe, les enseignants n'ont pas l'obligation de se faire vacciner et pourtant ils sont avec beaucoup d'enfants, donc il y a quand même des professions dans ce cette globalité du personnel soignant qui pourrait être remis au travail sans danger et tout le monde n'est pas ah au chevet de quelqu'un qui est en réanimation, il y a, il y a absolument aucune logique et aucun bon sens à à suspendre, quelqu'un qui ait du personnel administratif travaillant dans un établissement hospitalier, hospitalier au médico-social, je crois qu'il faut réfléchir à ça aussi, merci. Vraiment, monsieur le rapporteur, très peu de temps, parce que si vous voulez passer la nuit avec moi, il y a pas de souci. Mais en revanche, ce sera. à votre détriment, il a fallu. Il a fallu, madame la présidente, allez-y, il a fallu madame le président à tendre le jour de mon anniversaire que vous ayez des paroles aussi suave à mon oreille. Et je tiens à vous en remercier publiquement. Je voudrais simplement dire à notre excellente collègue que nous avons pensé au cas qu'elle vient de signaler, puisqu'il est prévu dans notre texte. les l'obligation vaccinale pourra être levé par catégorie successives de personnel effectivement la Haute autorité de santé pourra très bien dire que telle ou telle catégorie de personnel parce qu'elle est éloignée des personnes vulnérables, on peut lever son obligation vaccinale plutôt que pour d'autres.

à savoir comment est ce que nous faisons société ensemble et notre collègue Théophile là Dieu avec ses propres mots, mais nous ne sommes pas simplement sur une question à savoir combien de personnels soignants sont aujourd'hui interdits d'exercer leur profession est suspendu, nous ne sommes pas aujourd'hui à savoir quel est le ratio de personnes qui pourraient être des sapeurs pompiers qui ne le sont pas, nous sommes dans une question qui est, nous n'allons pas rouvrir le débat ici, je vous rassure, monsieur le Ministre, et mes collègues qui qui résulte de comment la gestion de cette crise sanitaire et de la situation vaccinale a été faite et discuter ici, au Parlement comme dans le reste de la société, donc, l'on pourrait se renvoyer autant que de besoin, qu'il s'agit d'un monde finalement marginal de personnes nous pourrions vous dire comme ça a été fait, qu'il y a un nombre très important de profession qui aujourd'hui sont en contact avec le public sont des vecteurs de transmission qui ont vécu cette 7ème vague à l'heure où les masques sont tombés, et qui pour autant n'étaient pas soumis à une obligation vaccinale et donc ce n'est pas simplement qu'une question anecdotique ou de décret à venir je crois que c'est très sincèrement aujourd'hui comment est-ce que certains se sont d'abord exclus à tort ou à raison, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit précédemment et comment est-ce que collectivement nous allons réintégrer l'ensemble de ces personnes pour continuer de faire société ensemble et de servir l'ensemble de la population, nous voterons bien évidemment notre amendement. Merci. Donc, nous allons procéder donc au scrutin public qui été demandée par le groupe, les républicains sur les amendements identiques 52 rectifié 60 rectifié, je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est défavorable, le scrutin public aura lieu dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin numéro 121 sur les amendements identiques numéro 52 rectifié quater et 60 rectifié compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs groupes politiques et à la présidence, nombre de votants 338 Nombre de suffrages exprimés 334 pour l'adoption 104 contre 230 le Sénat n'a pas. Adopté alors, nous passons à l'examen des amendements suivants le hein rectifier Madame Noël. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Comme évoqué tout à l'heure on amendement a pour objet de réintégrer immédiatement les soignants et d'abroger sans tarder cette obligation vaccinale, petite précision, mes chers collègues, lorsque je remets en cause le fait que le vaccin, puisse se protéger de la transmission et de de la portabilité du du du virus, je ne remets pas en cause son efficacité sur sa protection contre les formes graves, je me sens véritablement attaqué, à chaque fois et je pense que cette mise au point, elle est essentielle, regardons-nous, nous avons tous repris aujourd'hui une vie normale, on a plus de masque les gestes barrières, on les a un petit peu mis de côté, donc, oui, on est de nouveau dans une petite vague voilà de de d'épidémie de cas, mais encore une fois, ce ne sont pas forcément des cas graves et aujourd'hui le Covid il tue environ. j'ai regardé les derniers chiffres hein, ça se ça se tient, c'est entre 50 et 70 personnes par jour, sachez juste que le cancer tue entre 350 et 400 personnes par jour, on peut donc considérer qu'on est quand même rentré dans une phase endémique et que les conditions me semble aujourd'hui réunis, si elles ne sont pas réunies aujourd'hui quand le seront-elle, elle ne le seront jamais, parce que si on attend qu'il n'y ait plus de pression sur les hôpitaux, vu l'état dans lequel sont nos hôpitaux malheureusement on n'en sortira jamais, donc il faut quand même aussi se souvenir qu'il y a la quasi-totalité des pays dans le monde qui ont levé cette obligation vaccinale des soignants et ce qu'on va être le seul sur la planète à le maintenir. Bref, dans mon département, je tiens quand même à apporter mon témoignage, bon nombre de ces soignants et de pompiers sans perspective d'avenir ont d'ores et déjà opté pour une reconversion dans d'autres secteurs d'activité, ou alors dans certaines régions frontalières comme la Haute-Savoie, ils sont tout simplement partis en Suisse, il faut que cette obligation conclut n'est pas requise donc si vraiment je vous demande véritablement soutenir cet amendement merci monsieur le rapporteur. le nombre de morts du cancer au nombre de morts du Covid actuellement qu'il y a du point de vue de la vaccination des personnels une différence, c'est que on ne peut pas contaminé un malade du cancer, ou plutôt une personne en faisant qu'elles soient affectés par le cancer si on n'est pas vacciné, tandis qu'on peut éviter de contaminer malade de l'hôpital par le Covid si on n'est pas vacciné, c'est cette comparaison n'a pas tellement de sens, voilà ce que j'essaie d'expliquer à cette heure tardive de notre débat, en tout cas l'avis est défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, même avis madame la présidente merci alors pour explication de vote Monsieur Jomier. Oui, madame la présidente merci parce que, malgré l'heure tardive, on peut pas laisser dire dans cet hémicycle des choses qui sont totalement fausses. Hé oui parce que le vaccin n'annule pas la transmission mais la réduit et ça n'est pas rien : la réduction de la transmission, ça n'est pas inintéressant, on va le répéter à chaque fois. Que vous avancerait des des faits qui sont inexactes, mais nous ne sommes effectivement pas dans des dispositifs efficaces à 100 personne n'a prétendu que les vaccins éviter 100 pour des formes graves et 100 % des transmissions, c'est un outil, un parfait mais c'est le meilleur qu'on ait jusqu'à aujourd'hui, et puis deuxièmement il a tué ce virus depuis le début de l'année 25000 personnes. Sur les 6 premiers mois, ça fait pas 70 par jour, je vous invite à sortir votre calculette, ça fait 2 fois plus. Il tue, il a tué du 1er janvier au 30 juin on verra plus tard pour les chiffres du 17 juillet si ça vous amuse, mais 25000 personnes, ça veut dire une moyenne de 50000 par an et il en a tué cent cent il attend, lui et 150000 Français depuis le début de la l'épidémie, ça en fait un des problèmes de santé publique majeur de notre pays au même niveau que le tabac, l'alcool ou la pollution de l'air alors minimisé sans cesse les chiffres minimiser l'intérêt des outils de lutte, je me demande quel est le fond de tout ça. Qu'est-ce que vous poursuivez comme but de nier de nier la nécessité qu'une société adoptent des mécanismes collectifs pour se protéger contre une menace de sanitaire de premier ordre, hé ben moi, ça me laisse pantois parce que, hé oui, parce que vous faites simplement la défenseure du moi je, et je ne veux aucune contrainte et je balaye et je minimise sans cesse la réalité et vous ne pouvez pas le nier, c'est bien 50000 décès annuels sur la pente sur laquelle on est en ce moment.

faute de soignants faute de pompiers ont somme ces gens d'aller au travail, malade du Covid, enfin il faut quand même ici que quelqu'un le dise on les sommes d'aller travailler, parce qu'on a plus de personnel, oui, des infirmiers, des infirmières en réanimation, c'est pas la peine de de dîner des infirmiers et des infirmières en réanimation malade du Covid vont au chevet de leurs patients, il faut quand même que quelqu'un le dise ici, donc moi je voudrais savoir pourquoi se priver de ses personnels, franchement il vaut mieux qu'ils aillent travailler sans être malade, avec éventuellement un test PCR avant plutôt que des personnes vaccinées parce qu'ils sont vaccinés quand même travailler malade fiévreuse, enfin quand même il faut ouvrir les yeux, moi je ne sais pas je, je, je suis effaré de de cette discussion, je, je, j'attends, Monsieur le Ministre, votre réponse solennelle, dites-moi pourquoi vous acceptez que des personnels soignants et des sapeurs-pompiers soit obligé d'aller travailler alors qu'ils sont souffrant du Covid. merci madame la présidente, c'est pour soutenir Monsieur le Ministre, est Monsieur le Président l'amendement de Sylviane Noël également parce que il y a une chose que l'on sait aujourd'hui on essaie de prendre des décisions par rapport à la situation d'aujourd'hui, pas par rapport à la situation d'hier, on sait qu'aujourd'hui le le vaccin ne protège pas. En tout cas pas beaucoup de la de la contamination, première chose 2ème chose, on sait qu'il y a pas de hasard dans les grands nombres, il y a pas de hasard dans les grands nombres et à partir du moment où on sait très bien qu'il y a aujourd'hui énormément de contamination, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui énormément de soignants, de pompiers, d'autres personnes qui travaillent en ayant en ayant le Covid qui se sont d'ailleurs pas testé, y a, il y a effectivement une situation d'aujourd'hui qu'il faudrait prendre en compte parce que, entre quelqu'un qui est vaccinée malade du Covid qui travaille et quelqu'un qui ne peut pas travailler parce qu'il n'a pas été vacciné et quand on sait que cette vaccination ne protège pas, c'est peut-être le moment justement de, de, d'accélérer un peu sur le le retour des agents dans leur service au moment où on a le plus besoin et puis moi je pense pas franchement que ce soit une question de chiffres pour une question de nombre, c'est une question de principe dans la société, on peut peut-être se dire qu'à un moment donné, on les a exclus parce que on avait peut-être pas tous les éléments ont prêté de : fallait-il le faire à ce moment-là, mais si les éléments ont changé et ce qu'on laisse les citoyennes et les citoyens comme ça sur le bord de la route, dont un certain nombre de non plus de salaire depuis des mois et des mois alors qu'effectivement, je confirme ce qui vient d'être dit, d'autres citoyennes et citoyens qui sont malades et qui ont le Covid et vont travailler avec un masque, donc c'est aujourd'hui qu'il faut examiner la situation et c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut avancer, sans pour autant attendre que le gouvernement prenne une décision sous une autorité quelconque dont on ne sait pas d'ailleurs. Laquelle ce sera Merci madame la présidente, moi je voulais juste préciser que le taux de survie au Covid, c'est 99 8 % au pire, donc on ne parle pas d'une, on parle du pire 99 8 % de personnes survivent au Covid je voulais préciser aussi que si on pense que, au bout d'une 3e dose de vaccin, elle est valable 4 mois puisqu'au bout de 4 mois, il faut recommencer les, le personnel. Aujourd'hui dans quatre mois ne l'est plus, il n'est plus considéré comme avoir un schéma vaccinal complet donc, est-ce qu'on remet ce personnel en en cause, on sait que dans les hôpitaux aujourd'hui parce que il y a besoin de personnel, les chefs d'établissement n'oblige plus à la troisième ou à la 4ème dose sinon ils ont plus personne, donc c'est malhonnête, c'est malhonnête. Et peut-on, devons-nous rester dans dans une décision qui est aujourd'hui injuste et malhonnête. Merci monsieur opère. Merci madame la présidente, je le Ministre, mes chers collègues devant la mort, il faut être humble. Devant la maladie, il faut être humble, arrêtons de nous battre avec des chiffres, nous sommes face à une injustice à une inégalité. Face à des gens qui n'ont plus de travail. Qui n'ont pas la possibilité. Puisqu'ils sont toujours intégrés, d'aller chercher un autre travail. Un peu d'humanité. Hospital, l'hôpital, ça veut dire, ça vient d'hospitalité, un peu d'hospitalité. Merci, alors je mets Monsieur Monsieur air oui monsieur l'air ça vous. J'entends parler d'humilité, je crois qu'il en faut un petit peu d'humilité, effectivement j'entends parler aussi de principe, je crois qu'il en faut des principes, on a vraiment un problème dans notre société, de respect, d'autorité, il y a un manque d'autorité, alors je ne parle pas de l'autoritarisme, les choses, mais d'une autorité de compétence, alors on peut dire que l'Académie de médecine, ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi, les facultés de médecine, c'est n'importe quoi, no haute autorité de la santé, c'est n'importe quoi, on peut citer un professeur moi je pourrais citer le professeur Raoult aussi bien qui était une sommité faut arrêter, je pense que dans une société dans notre République, qui prône aussi la solidarité, la, la fraternité, faut avoir respect de certaines règles, si on respecte pas un minimum de règles, si on ne les fait pas respectée si on n'est pas exemplaire, quelle image on donne à l'ensemble de notre société à nos enfants au simple citoyens qui font confiance lorsqu'ils vont dans des services de soins pour recevoir justement des soins qui sont peut-être pas exactement qui sont peut-être pas exactement ce que l'on souhaiterait mais qui, qui sont l'objet de consensus le le fruit de consensus scientifique et qui ont été approuvées effectivement un peu d'humidité, s'il vous plaît, et puis un respect de certains principes qui est celui du respect de l'autorité. Merci. Alors je mets je mets aux voix l'amendement numéro 1, rectifier, qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour.

les personnels aujourd'hui suspendu, n'ont pas vocation à le rester ad eternam. Ils ont bien vocation à réintégrer leur travail, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté la suppression de cet article 2 bis, en revanche, moi j'ai un autre problème si le contrat de travail n'est pas suspendu, j'ai un problème moi d'affectation et j'ai un problème de respect et de discipline d'autorité évoqué il y a un moment de de discipline quelque part, oui à la réintégration mais non à l'affectation au chevet des malades et c'est la raison pour laquelle je propose de moyen terme de dire si cette vocation, hé bien là ils peuvent réintégrer leur sud d'accord pour heure la réintégration mais non pas à leur affectation du malade ou des personnes fragiles ou vulnérables,

et je parle sous votre contrôle, qu'il y a 72 métiers éligibles à l'obligation vaccinale il y a une seule non, c'est une vocation plus que professionnel éthique, elle est morale, c'est de dire que vous devez prendre soin de vos patients et donc moi je propose que, au lieu de laisser à la seule discrétion du gouvernement, on peut faire confiance ou de laisser à une autre autorité de santé ou je ne sais quel autre machin, quelle que soit leur expertise quand c'est au législateur de dire à ce cette autorité réglementaire que oui, d'ores et déjà, nous respectons cette autorité-là nous respectons cette morale, hein, et que nous excluons une affectation au chevet du mal, a-t-elle et le sens de l'amendement qui vous est présenté.

J'aimerais comprendre l'explication : en quoi le pouvoir dans directeur c'est de diminuer, il lui serait impossible, puisque le contrat de travail n'est pas rompu de réaffecter en quoi. En quoi il est ça permettrait aux gens de retrouver leur travail. En quoi c'est impossible chez moi, avoir une explication plus claire bon, OK, je j'ai compris, il faut aller vite, mais moi je ne me pose pas la réintégration je m'oppose à une affectation du malade. je mets aux voix donc l'amendement trente-cinq il a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour, qui est contre qui s'abstient. Non pas adopté l'amendement 16 Monsieur Le Carré. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors cet amendement qu'on vous pourrez considéré comme un amendement de repli après le rejet des différents amendements, notamment de l'amendement de de Sylvie Noël c'est un amendement qui ne se pose : qui ne se situe place pas sur le le débat de l'obligation vaccinale des soignants qui ne remet pas en cause la rédaction proposée par notre rapporteur et la Commission, mais qui. Parce que la situation actuelle l'exige, parce que notre département la Haute-Savoie et dans une situation sanitaire ou l'aspirateur de ressources humaines vers la Suisse est déjà extrêmement puissants cette interdiction faite aux soignants d'exercer leur métier en France, les conduit directement vers des employeurs suisses. Parce que cette règle là n'existe pas, n'existe plus en Suisse et que cette réalité, elle est transposable dans tout un tas de de de département à Besançon dans 10 grandes agglomérations dans le monde rural, moi je pense que le temps est venu de la réintégration immédiate des soignants, donc je touche pas à l'obligation vaccinale on touche pas à la rédaction du rapporteur Philippe Bas, mais de manière mécanique et juridique, cet amendement permet dès la promulgation de la loi que les soignants non vaccinés ou qui ne sont pas à jour de leurs obligations vaccinales sont réintégrés, ça permet de dépassionner le débat, d'être plus juridique mais je pense que maintenant le temps est venu, le débat a été utile, je crois qu'il était utile et merci, monsieur le rapporteur de l'avoir permis, j'espère, Monsieur le Ministre, que si vous ne réintégrait pas les soignants non vaccinés que vous aurez que vous arriverez dans les mois qui viennent, à trouver un argumentaire un véhicule législatif pour le faire. Merci, alors l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Malgré l'ingéniosité de cet amendement et peut être à cause de cette ingéniosité, la commission a émis un avis défavorable. Merci la vie de du gouvernement Monsieur le Ministre, même avis madame la présidente, merci. Alors j'ai été

j'ai été saisi d'une demande de scrutin public à par le groupe, les républicains sur l'article 2 bis, donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

as du scrutin numéro 122 sur l'article numéro 2 bis, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs groupes politiques et notifié à la présidence, nombre de votants 339 nombre de suffrages exprimés 319 pour l'adoption 229 contre 90, le Sénat a adopté. Alors 3 amendements après la. C'est que le bis qui font l'objet d'une discussion commune. Alors le 63 Madame Cohen de poursuivre notre chemin en en proposant donc un amendement on, on dit que pour permettre la continuité de la prise en charge des patients et et pallier notamment les urgences qui sont réels, du fait de la situation dramatique que nous vivons ne manque de personnel, de fermetures de lits et cetera, même si c'est pas la radiation, la suspension des personnels qui en est là, la cause nous demandons donc leur leur réintégration, l'amendement 63 rectifier et je vais vous faire gagner du temps, madame la présidente, je vais proposer le soixante-neuf rectifié bis, si vous me le permettez tout aussi rapidement, c'est un amendement donc de repli et nous proposons également la réintégration de ce personnel mais en imposant une condition et cette condition c'est de justifier d'un test virologique négatif à chaque prise de service, donc c'est aussi une ouverture, merci madame la présidente.

Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, alors en plus des soignants hospitaliers, il y a environ 1350 professionnels de santé libéraux, des médecins, des kinésithérapeutes, des cardiologues, des gynécologues, et caetera, qui sont interdits d'exercer pour le non respect de l'obligation vaccinale, selon les chiffres donnés par l'assurance maladie en novembre 2021 alors que les zones qualifiées de déserts médicaux augmentent, y compris dans les grandes villes, il est urgent de supprimer cette obligation vaccinale dont on connaît maintenant les limites, s'agissant de la transmission du virus à tout cela, ça ne suffit pas encore et pour décourager encore ces professions médicales qui manquent cruellement de candidats, hé bien depuis quelques semaines, on assiste à une véritable pratique de chasse aux médecins, organisée par les directions régionales du service médical ou par les caisses primaires d'assurance maladie en effet celle-ci signale à l'Ordre des médecins, les praticiens et les mettent, mettent en cause leurs prescriptions et les Liens qu'ils ont avec leurs patients, ils sont convoqués devant des pseudo tribunal tribunaux pardon sont l'objet de représailles sont suspendu ou sanctionné par des interdictions d'exercer jusqu'où irons-nous, nous avons besoin de tous nos médecins et des médecins libéraux aussi, et les médecins sont là pour soigner et non pas pour être sanctionné. Merci,

il est un peu plus de 2 ans, du jour au lendemain, les soignants et assimilés comme les pompiers ont dû s'adapter pour tenter de contrer ce nouveau virus qui était la Covid 19 nous étions alors en guerre et tous ont répondu présents, les Français chaque soir applaudissait leur héros entre-temps le gouvernement établissait une liste de professions soumises à l'obligation vaccinale, aujourd'hui, la plupart d'entre nous avons repris une vie normale face à ce virus, et pourtant les pompiers demeure soumis à cette obligation vaccinale, alors même que nous savons que la vaccination n'empêche pas la transmission du virus, alors même que dans nos territoires touchés par la désertification médicale un pompier volontaire non vaccinés, peut faire la différence dans la prise en charge d'une urgence vitale, alors même que nous sommes les témoins d'incendie d'une exceptionnelle force qui ravage certains de nos territoires. Aujourd'hui, le gouvernement continue donc de préférer de rappeler des personnels vacciné mais malade du Covid que de faire appel à des professionnels non vaccinés négatif, cessons d'avoir une vision punitive et ayons une réflexion pragmatique, on parle ici de 140 pompiers professionnels et de 5000 sapeurs-pompiers volontaires, cet amendement visant à supprimer l'obligation vaccinale pour les pompiers et ainsi permettre à tous d'être utile et d'être sur le terrain pour répondre à leur vocation première : protéger les biens et secourir les victimes. Merci, alors l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Sur l'amendement 63 rectifier bis, l'avis de la commission est défavorable, c'est un amendement qui prévoit que les directeurs réintègre c'est-à-dire doivent le faire, les personnels soumis à l'obligation vaccinale sur l'amendement 69 rectifié la vie est également défavorable cet amendement pour sa souche prévoit que les directeurs non pas réintègre mais peuvent réintégrer les personnels soumis à l'obligation vaccinale qui ne sont pas vaccinés, et les 2 amendements sous-amendements sont également rejetés par la commission des lois, le premier, le 23 rectifié bis parce qu'il exonère les médecins libéraux de l'obligation vaccinale est le suivant : de notre collègue Christian Klinger, parce qu'il dit que les pompiers n'ont pas non plus d'obligation vaccinale désormais, c'est beaucoup trop général : alors, chers collègues, s'agissant des pompiers, on n'a pas suffisamment parlé ce soir et je crois que il était important que votre abonnement soit là pour nous donner l'occasion de le faire, mais à ma connaissance, il n'y aurait que entre 100 et 200 pompiers pour toute la France, qui aurait refusé de se faire vacciner si vous voulez démentir ce chiffre nous effectivement une information que je n'ai pas pu trouver, j'ai en réalité des informations qui proviennent de sources syndicales, je reconnais qu'elles ne sont pas d'une fiabilité totale mais peut-être avez-vous mieux à proposer, en tous les cas, je ne crois pas que nous soyons privés de nombreux sapeurs-pompiers pour faire face aux urgences du moment, et notamment à ces terribles incendies de forêt de la Gironde et de la Bretagne, voilà pourquoi les les avis de la commission sont défavorables à ces amendements et sous-amendements. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, même avis madame la présidente, merci. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement 63 que reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour.

Madame la présidente, merci monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, alors l'article 3, demandent au gouvernement une évaluation du cadre juridique en vigueur pour lutter contre les pandémies sans avoir recours à un régime d'exception ce cadre juridique est essentiel pour ne plus recourir à des mesures d'état d'urgence, mais il devra aussi s'étendre à une évaluation des décisions médicales et sanitaires après 2 ans d'absence totale de transparence sur les expertises qui ont défini la stratégie de vaccination l'opacité continue sur le sujet des effets indésirables en effet 25 % d'effets indésirables graves sont confirmés par l'ANSM. Ce qui est beaucoup plus que tout autre traitement ou vaccin normalement on aurait suspendu la prescription ou la vente de tels traitements à ce sujet, je veux revenir sur la question que j'ai posée lors des éditions des auditions de l'OPA, c'était en mai dernier au Sénat concernant la vaccination de 22490 enfants de 0 à 12 ans, et notamment de 4512 enfants de 0 à 4 ans hors autorisation et avec des doses adultes parmi eux des enfants de moins de 5 ans 4512 avec une dose et 2435 avec de 12 110 puissent disposer d'études cliniques ni d'autorisation légale, l'ANSM. Répond qu'elle réceptionne tous les signaux envoyés sans distinction d'âge ou de situation et que toute déclaration et suivi certes mais tout effet secondaire a-t-il été déclaré comment cette cohorte d'enfants et tel suivie fait-elle l'objet d'un suivi spécifique et pourquoi ce régime d'exception sur cette cohorte, que peut-on me répondre à ce sujet, merci. Merci madame Angèle Préville. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, plus de 2 ans après le début de la pandémie, le constat est quelque part Gramat dramatique, il y a eu 150000 morts et comme le rappelait mon collègue Bernard Jomier au rythme de certainement 50000 morts par an. Et. Ceux-là sans qu'une certaine forme de cérémonie ou d'hommage national qui aurait pu être une initiative d'autant plus que nombreux sont nos concitoyens affectés d'autant plus qu'il a été parfois qui ont été parfois dans l'impossibilité de vivre ces deuil dignement, notamment au début de la pandémie, malheureusement, d'autres souffrances touche certains de nos concitoyens, à savoir le Covid long, il s'agit d'une particularité spécifique au Covid 19, nous n'avons jamais connu ça, avant, nous sommes devant une situation inédite et visiblement, nous n'avons ni le suivi ni l'accompagnement adapté à cette affection de longue durée qui déjoue tous les schémas habituels, j'ai été interpellé par des concitoyens qui vivent des situations d'impasse de véritables errance médicale au bout d'un suivi qui avait pourtant bien commencé, mis en place, mais qui s'arrête, d'une certaine manière, brutalement, car il n'a pas été tenu compte du caractère très particulier de ces affections qui sont d'une grande complexité qui nécessite plus de temps de prise en charge déjà qui présente une multitude de symptômes différents et des thérapies qui ne sont pas encore cristallisées, il faudra sans doute du temps en tout état de cause, je déplore que l'amendement que j'avais déposé qui demandait un rapport et qui a été déclarée recevable sur ce sujet-là sur l'évolution et la prise en charge et diverses mesures mises en place pour l'accompagnement de ces Covid long n'ait pas été n'ait pas pu être examiné ce soir j'ai bien vu qu'il avait une feuille de route Publié le 17 mars 2022, mais j'ai cru comprendre que certaines de ces dispositions ne serait pas appliquée car j'ai dans mon département des comme je le disais tout à l'heure des des patients qui sont en déshérence totale est complètement des chers. Merci. Madame Victoire Jasmin. merci madame la présidente, monsieur le Ministre je voudrais à ce stade, attirer votre attention sur les conséquences de certaines des mesures qui ont été prises. Il y a un centre de radiologie aux Abymes, en Guadeloupe, un des rares parce qu'elle n'a pas tant que ça, qui est fermé, avec l'ensemble de son personnel et cela pose un véritable problème pour la prévention, concernant les cancers du sein parce que c'est un centre qui faisait une bonne partie des dépistages concernant le le cancer du sein, donc en Guadeloupe il y a de grandes difficultés parce que des certaines conséquences de ces fermetures d'entreprises, parce qu'il suffit, il suffit d'un. Après les modalités de cette mise en place de, de, de, du texte du mois de d'août dernier, hé bien. Il se trouve que les patrons quand ils ne sont pas vaccinés, hé bien c'est toute l'entreprise qui ferme, voilà donc le centre de radiologie à du gaz 11 fermée et ce sont les épices dépistages qui sont vraiment en grande difficulté, les femmes en particulier. Merci, alors nous allons passer l'examen de l'amendement numéro 10 à Monsieur Bénard Roche. Merci madame la présidente, la loi du 11 mai 2020 de prorogation de l'état d'urgence sanitaire a autorisé la création temporaire de de fichier de traitement de données à caractère personnel les fichiers Sidep et contact Covid la centralisation et la consultation de ses données de santé contenant plusieurs mention à caractère personnel on fait partie intégrante de la gestion de l'épidémie, ces 2 dernières années, ces fichiers ont été maintes fois prorogé sans que nous ayons pu évaluer la pacte effectif de ces fichiers de traçage sur la stratégie sanitaire globale, les auteurs du présent amendement demande donc à ce qu'une évaluation du cadre juridique de ces fichiers soit réalisée afin de définir, notamment si les protections constitutionnelles et conventionnelles du droit au respect de la vie privée sont respectées et s'il y a un risque de pérennisation de ces outils de traçage de la population dans notre droit commun. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, monsieur ben arrogent s'est montré aussi convaincant cet après-midi devant la commission que ce soir devant l'hémicycle, c'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis favorable. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, même avis madame la présidente, merci. Donc je mets aux voix l'amendement numéro 10, qui a reçu un avis favorable de la commission et du gouvernement. Donc, il est pour.

Madame la présidente, le présent amendement a pour objet de rétablir l'article IV du présent projet de loi adopté en commission à l'Assemblée nationale. Et qui avait pour objet d'enjoindre le gouvernement a présenté au Parlement un rapport d'analyse de l'efficacité et de coût des mesures prises par le gouvernement sur la propagation de l'épidémie, ainsi que leur Zapa acte sur le système de santé sur l'état de santé de la population sur l'adhésion de la population à la vaccination à la Covid dix et sur l'état général de l'économie et des finances publiques, après plus de 2 ans de gestion de l'épidémie de Covid 19 ils sont fondamentales d'établir un bilan sur l'efficacité et le coût des mesures prises dans ce contexte d'autant plus qu'un autre grand regret, le Parlement n'a été que trop peu associés à ces décisions, bien sûr, l'argument des hausses, texte que nous avons voté ne pèse en fait pas grand chose face au refus systématique de partage des informations, en particulier les avis et les notes du conseil scientifique ni face à la volonté du gouvernement de ne pas intégrer des propositions qui n'étaient pas issus du gouvernement, il est plus que temps d'en faire rendre des côtes de permettre, en transparence de faire véritables retour d'expérience et de mesurer avec lucidité et humilité, les mesures que ce gouvernement a porté lors de sa gestion de la crise sanitaire de déterminer celles qui été bénéfique de quantifier ces bénéfices, celle qu'il aurait été, dans une moindre mesure, voire de pointer les erreurs commises, comme celle par exemple de la gestion des masques que récemment une décision du Conseil d'État a mis en avant dans la prise en compte des spécificités territoriales ou la consultation des élus locaux, bilan présenté devant le Parlement, semble également tout à fait nécessaire au vu de la persistance de l'épidémie de Covid 19 de son caractère épisodique et du développement de ces variants. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. L'avis est défavorable, merci l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, ces messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, votre amendement vise à prévoir un rapport exposant les mesures prises par le gouvernement aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid 19 et qui analyserait l'efficacité le coup et plusieurs des impacts de ces mesures, si ce rapport était présent dans la version adoptée par l'Assemblée nationale, il ne figure plus actuellement dans le texte adopté par votre commission des lois. Il est vrai que plusieurs rapports ont d'ores et déjà été portés à l'attention du Parlement sur les mesures de gestion de crise sanitaire en présentant un bilan de l'application de ces mesures, conformément à ce qui était prévu par la loi. Cela étant, je m'en remets à la sagesse de votre assemblée pour déterminer la nécessité d'un tel, rapport. Merci donc Alors je mets aux voix donc l'amendement numéro 8 qui a reçu un avis défavorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient pas adopté alors l'amendement 47 rectifie Madame Conway Mouret. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre amendement demande au gouvernement un rapport alors je sais que c'est pas la demande la plus populaire, mais j'espère que mon argumentaire vous convaincra du bien-fondé de la demande qui permettrait au Parlement, non seulement d'avoir une vision globale des diverses mesures qui ont été prises à destination des Français établis hors de France depuis le déclenchement de la crise sanitaire, mais surtout de tirer les leçons de leur efficacité dans le souci d'améliorer ce qui a été mise en place et d'éviter de reproduire les erreurs cette pandémie obliger tous les États à prendre des mesures sans pouvoir en évaluer toutes les conséquences, puisque la situation était inédite, heures et demie plus tard, le temps est venu d'effectuer un retour d'expérience afin d'être à même d'anticiper et de nous préparer aux crises à venir et, malheureusement, je crains qu'elle ne soient nombreuses, sur le plan sanitaire de nombreux Français résidant à l'étranger en particulier hors de l'espace Schengen sont restés dans le flou pendant de longs mois, exigence d'un motif impérieux pour entrer en France, finalement annulée par le Conseil d'État non reconnaissance des QR codes délivré par leur pays de résidence difficulté parfois à trouver sur place un vaccin reconnu par l'Europe sur vaccination pour être en conformité avec le droit local et loi de français jusqu'à 5 ou 6 injections en un an, pour certaines personnes au au-delà, ce sont tous les pans de la vie de nos compatriotes qui ont été impactés pour les aider, des moyens importants ont été engagés et des aides ont été alloués, bien que tous les crédits n'est pas toujours été dépensés feu a aussi soutenu son réseau et accompagner les familles toutefois les critères d'accès aux aides sociales, se sont avérés très restrictif de multiples entreprises françaises n'ont pas pu se relever se sont vus dans la capacité de s'acquitter des frais de scolarité conséquemment à la perte de leur emploi et de leurs revenus, nos instituts et nos alliances françaises ont souffert, tout comme nos postes diplomatiques et consulaires quant accumulé du retard entravant encore aujourd'hui les démarches administratives essentielle de nos concitoyens, nous avons fait de nombreuses interventions qui sont restées jusqu'alors sans réponse pense que un rapport exhaustif nous éviterait pléthore de courrier et de questions à venir au concours qui rassemblerait ainsi. L'ensemble des données on madame la présidente, merci beaucoup, l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. La Commission comme vous le savez très attentive à la situation des Français de l'étranger, c'est la raison pour laquelle elle a examiné avec beaucoup de réflexions, cet amendement mais il nous a paru poser un problème de principe, chers collègues, c'est que l'évaluation des politiques publiques, c'est une prérogative constitutionnelle essentiel du Parlement. Et la déléguée au gouvernement en lui demandant un rapport d'évaluation d'une politique publique, ça nous paraît être un renoncement pour nous, je crois qu'il vaudrait beaucoup mieux qu'au sein des commissions compétentes vous plaignez la même cause et que nous nous en parlions de cette question que vous soulevez à juste titre, de l'évaluation de l'efficacité et de l'impact, et du coup dans les différents domaines que vous citez de la lutte contre le Covid en ce qui concerne naturellement les Français de l'étranger, donc, voyons les choses très clairement, faisons en sorte que le Sénat assume ses responsabilités, sans les délégués au gouvernement : avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Le gouvernement s'en remet à la sagesse de votre out à son. Merci beaucoup, donc je mets aux voix l'amendement 47. dis si Monsieur Lurel. Si vous faites court ce sera pas. Ah, ce serait très court et en plus c'est un gros sujet, madame la présidente, je profite à la faveur de l'examen de la bonne pour collègues pour adresser une demande et pour pour voir une supplique au au ministère de la Santé, personne ne sait qu'le nombre de suspendu de soignants suspendus en Guadeloupe, en mai dernier, l'ARS a publié un chiffre qui n'est pas vérifié 631 suspendu. Et à peu près une centaine qui n'aurait pas fait de choix et qui serait aujourd'hui suspendu, pourriez-vous demander à votre ARS de publier des chiffres clairs et puis d'avoir la pédagogie de la communication, s'il vous plaît, je le dis pour que vous l'entendiez et que vous passiez les instructions merci. Merci. Alors donc je mets aux voix l'amendement 47 qui a reçu un avis défavorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Ces contrats. Qui s'abstient n'est pas s'adopté l'amendement 24 de Madame Müller Bronn. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, à heure à travers cet amendement, il s'agit de demander dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport que le gouvernement présente devant le Parlement, consolider sur les effets indésirables des vaccins contre la Covid 19 incluant une comparaison avec les vaccins contre la grippe, ce rapport répond à l'obligation inscrite dans l'article R 41 27 tiré 35 du code de la santé publique qui prévoit que le corps médical doit au patient une information loyale approprie appropriée sur son état, les investigations et les soins qui lui propose, il répond également au principe de consentement éclairé consacrés par le code de Nuremberg en 1947 en présence d'un risque inconnu et d'une technique vaccinal, toujours en phase d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle dont les études n'inclut pas la troisième et la quatrième, comme le souligne le rapport d'étape de l'OPS l'Opecst pardon, merci, publié le 9 juin 2022 sur les effets indésirables des vaccins contre la Covid 19 et le système de pharmacovigilance une communication transparente et complète est nécessaire sur l'existence d'effets indésirables, ainsi qu'une action vigoureuse pour encourager les professionnels de santé, a déclaré des événements indésirables, mais aussi un soutien adapté au système de pharmacovigilance dans son ensemble pour garantir les conditions de la confiance des citoyens dans la capacité des autorités sanitaires à assurer leur sécurité. Merci, à travers cet amendement à compter de la promulgation de la présente loi et afin de procéder à une analyse de la mortalité toutes causes confondues, en fonction du statut vaccinal des personnes, les données du système national de données de santé sont rendus accessibles de manière anonymisé à la recherche scientifique pour l'ensemble de ces acteurs en effet en moyenne 70 % des personnes entrées à l'hôpital et déclaré Covid sont vaccinés, ce sont les chiffres de l'adresse qui sont en accès libre, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques qui dépend des ministères de la Santé et des finances, mais il serait intéressant d'en connaître beaucoup plus l'âge, le sexe des personnes, les dates de vaccination, les marques et les numéros de lots de vaccins utilisés les dates d'injection afin de bénéficier d'un référentiel de comparaison et enfin la date de décès des personnes toutes ces données existent dans le système national des données de santé, mais elles ne sont pas accessibles en toute transparence, à la recherche scientifique, voilà l'objet de cet amendement, il servirait de preuve définitive de causalité. Et viendrait appuyer les remontées de pharmacovigilance. Merci, sur l'amendement numéro 24 l'avis de la commission est défavorable et là justement, on est déjà dans les travaux pratiques, vous les avez-vous même cité l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques est en train de faire le travail, faisons-lui confiance, il incarne justement la responsabilité, la mission d'évaluation des politiques publiques du Parlement n'abdique ont pas de nos propres responsabilités en demandant des rapports que d'ailleurs il faut le dire, le gouvernement n'ait jamais tenu de produire, même quand tu nous avons voté la demande d'un rapport, mais nous n'avons pas le droit de faire des injonctions au gouvernement, en revanche, nous avons le droit et même le devoir d'évaluer les politiques publiques et s'agissant de votre 2ème amendement c'est le vingt-cinq il concerne l'accès des chercheurs au système national des données de santé sur la mortalité relative au statut vaccinal mais en vérité, cet amendement est satisfait par le droit en vigueur, c'est le 6ème de l'article L. 1 du code de la santé publique, c'est la raison pour laquelle je vous demanderai de retirer ce 2ème amendement sinon de la commission a émis un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, même avis madame la présidente, merci. Si beaucoup donc je mets aux voix l'amendement 24 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour.

Non mais Madame Müller Bronn je je lance voilà et on a les avis donc le vingt-quatre défavorable de la Commission et du gouvernement, donc qui est pour, qui est contrat qui s'abstient

passons à l'amendement 59 même Cohen. à la limitation des déplacements en passant par un couvre-feu le soir, mais à aucun moment, ce même gouvernement n'est revenu sur les origines du problème : le manque de lits d'hospitalisation dans notre pays et la pénurie du personnel soignant, pire, il y a eu une politique qui a consisté à fermer des des lits pendant cette crise sanitaire 5700 en pleine pandémie et 17000 lits d'hospitalisation depuis l'élection du président Macron en 2017 après l'alerte, fin mai, de 120 services d'urgence, le président de la République a confié à monsieur le ministre de la Santé, pas encore ministre à l'époque, la réalisation d'un rapport flash sur les urgences, ce rapport à formuler 41 préconisations mais malheureusement aucune n'a suggéré de tirer les conséquences des fermetures de lits d'hôpitaux en France, due notamment au manque de moyens, c'est ce que nous demandons une nouvelle fois aujourd'hui avec cet amendement, nous savons bien, ces fermetures de lits d'hôpitaux s'inscrive dans une cohérence et une logique gestionnaire qui dépasse la simple question de la pandémie et de ce dernier quinquennat bien que celui-ci et empirer la situation, nous avons donc besoin plus que jamais de pouvoir tirer un bilan de cette politique, l'argument opposable de ne pas voter des rapports de la commission ne tiendrait pas puisque notre haute assemblée avait voté la remise de ce rapport en juillet dernier et nous en étions très satisfait et là, cet amendement a terminé sa course prématurément en commission mixte paritaire, nous comptons cette fois-ci sur le rapport de force favorable au Sénat pour que cet amendement, une fois votée dépasse le stade de la CMP et soit définitivement adopté afin de faire évoluer les choses et d'enrayer les rouages du sacro-saint lean management que le gouvernement entend poursuivre dans la gestion de notre système hospitalier. Public

Non, je veux bien que leur leur soit tardive ou ou au contraire si qu'il soit très tôt, mais on est en train de parler quand même d'un d'un sujet qui est extrêmement préoccupant, on peut changer d'avis, effectivement, mais je ne comprends pas pourquoi majoritairement notre haute assemblée avait trouvé juste et efficace d'avoir la possibilité d'avoir ce bilan de pouvoir mesurer les conséquences des fermetures incessantes de lits d'hospitalisation qui se poursuivent aujourd'hui et nous sommes alertés par les personnels soignants et là

de bilan alors qu'il y a quelques mois, on était prêt, ensemble, à avoir ces données, il me semble que quand on fait des choix politiques, il est extrêmement important d'en mesurer les conséquences et d'avoir des données précises, c'est ce que nous demandons au travers d'un rapport, ils ne vont pas aller plus loin, compte tenu effectivement des contraintes qui nous sont hein vous le savez très bien monsieur le rapporteur. Merci. Qui alors je vais mettre aux voix l'amendement 59 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est donc pas adoptée et comme vous aimez les rapports, je vous conseille l'excellent rapport qui vient de sortir sur l'application des lois, où vous pourrez retrouver justement le taux de du nombre de rapports qui sont effectués par le gouvernement, y compris sur les rapports des gouvernements mais je vous laisse le livre est intéressant.

madame la présidente, monsieur le Ministre, chers collègues, à cette heure tardive, je voulais saluer la sagesse, la modération, la prudence et le réalisme du gouvernement qui a parlé de veille et sécurité sanitaire, finalement, c'est assez clair, alors monsieur le rapporteur, a voulu faire un peu de zèle une peu permettra de le dire en nous proposant, projet de loi mettant fin au régime d'exception par pour lutter contre l'épidémie, le seul problème c'est que ça ne met pas tout à fait enfin au régime d'exception puisque il reste le si DEP, il reste le contact Covid ainsi que le Pass Frontières et quelques autres choses, donc nous pensons que c'est finalement plus réaliste d'en revenir au tête au titre du gouvernement, mais enfin on ne va pas passer la nuit là dessus, mes chers collègues. Si l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, le sujet d'une grande importance symbolique, il mérite bien qu'on passe, chers collègues, un moment pour en discuter, je suis sûr que les autres collègues de l'hémicycle apprécieront ce débat entre questeur. Je voudrais vous dire sur collègue s'agissant des titres des projets de loi et des propositions de loi d'ailleurs. Qu'on pourrait écrire des romans avec. Mais qu'il vaut mieux ne pas le faire, car ce serait souvent des romans triste. S'agissant du titre qui avait retenu le gouvernement, je crois qu'il ne disait pas l'essentiel, s'agissant du titre que la commission des lois adoptées, je crois qu'il ne couvre pas de manière exhaustive la totalité des articles du texte, il est vrai qu'aucun titre ne peut couvrir de manière exhaustive toutes les dispositions d'un texte, il doit donc se concentrer sur ce qui est fondamental, ce qui est fondamental et qui résulte d'ailleurs du travail que nous avons conduit ensemble sur tous les bancs, cet après-midi et ce soir c'est que. Si ce texte est adopté à la suite d'un accord en commission mixte paritaire promulguée par le président de la République. Dès le jour de sa promulgation. C'est la liberté retrouvée pour les Français. La confiance dans leur esprit de responsabilité pour limiter les risques de contamination. Le retour à l'état du droit d'avant le Covid la fermeture d'une parenthèse. Il a bien a fallu accepter de l'ouvrir cette parenthèse mais elle sera fermée et il ne reste plus à titre résiduel et virtuel que. 2 dispositions permettant de faire face pendant quelques mois encore. Ah, l'irruption d'un problème majeur. Sans pouvoir établir le jamais le Pass le Pass vaccinal le Pass sanitaire le confinement, le couvre-feu, l'interdiction de réunion publique, l'interdiction de rassemblement et de manifestations, l'interdiction de sortir sans masque. Voilà la réalité et donc c'est simplement par honnêteté intellectuelle, compte tenu de ce qu'est la nature même de ce texte, une fois transformé en profondeur par le Sénat, que nous avons décidé de vous proposer mais la commission des Lois proposent le Sénat dispose que nous avons décidé de vous proposer de changer le titre pour dire qu'il met fin à cette période d'exception et qu'on rentre maintenant et nous étions impatients, que ce soit le quinze jours dans. Le droit commun, c'est très important. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. ça, madame la présidente. Merci, alors je mise aux voix, donc l'amendement cinquante, qui a reçu un avis défavorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour,

Si madame la présidente, nous avons besoin, mais monsieur, madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous avons besoin de contrôler les voyageurs, nous avons besoin de poursuivants les vaccinations, du reste, les vaccinations qui ont très peu d'effets secondaires et ça va être l'heure de la 4ème dose pour que notre pays puisse poursuivre on la vie avec le Covid et ses variants sans que les hôpitaux les réanimations soit submergés avec des Epad sécurisé et notre économie maintenue alors bon, j'aurais souhaité que mon amendement, avec la possibilité de présentation pour les voyageurs de l'un des 3 documents du Pass sanitaire je rappelle test Covid vaccin rétablissement selon le droit européen soit accepté et favoriser la vaccination, nous aurions souhaité aussi que l'HAS dans l'article 2 bis informe éclairent le gouvernement qui devrait, à notre sens décidé mais bien sûr, l'important, c'était quand même de rétablir l'article de même avec un seul test Covid et je suppose que l'HAS prendra des décisions en synergie avec le gouvernement en ce qui me concerne, donc je voterai ce projet de loi et les sénateurs mon groupe s'abstiendront merci. Merci, je vous indique simplement qu'il y aura un scrutin public a demandé par le groupe, les républicains sur l'ensemble du texte monsieur Bénard Roche. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente, notre groupe s'abstiendra sur ce texte, certes, un certain nombre d'avancées, par exemple sur le le le positionnement dans le texte d'une réelle abrogation de l'état d'urgence sanitaire exprimé clairement à l'article là le début de de la fixation de quatre juridique sur une possible fait de suspensions de soignants ou l'obligation de repasser devant le Parlement, au bout d'un mois nous paraissent gracios de la réintroduction de certificat de voyage limitée à la présentation de tests négatifs et ce y compris pour les mineurs ne nous pas repas équilibrés, les critères même pour réinstaurer des restrictions, nous sommes trop flou et là c'une fois de plus trop de marge d'appréciation au gouvernement, nous n'avons pas oublié les tergiversations du gouvernement face aux variants brésiliens, nous n'avons pas oublié la sourde oreille face aux demandes des élus corses, au moment de le ou leurs hôpitaux et c'est saturé, nous n'avons pas oublier les mesures différenciées, qui avait été prise par exemple entre le TER et le TGV, l'absence de critères objectifs de mise en place de restrictions aussi importante que celle d'aller et venir vont contre nos idées de dialogue poussées entre l'exécutif et le législatif, car nous savons légiférer vite vous 12, il avait déjà forcé, Monsieur le Ministre, donc l'excuse de l'urgence ne nous convient pas, de manière plus grave ce texte vous présenterez sur la qualité de l'air en prévision, par exemple de la rentrée, rien sur l'encadrement des masques du rien sur l'avenir de la campagne de vaccination qui, pour le 2ème rappel est vraiment à la traîne, rien sur la gratuité élargi de test PCR obligatoires aussi, nous nous abstiendrons à regret de n'avoir pu au moins discuter d'un certain nombre de mesures que dans le groupe a pu proposer depuis près de 2 ans et que certaines décisions d'irrecevabilité nous empêché de défendre ici. Merci monsieur le castor sueur. Oui. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour nous, il y a un point central, c'est que l'article de soit rétablie, c'est une question de responsabilité, il était irresponsable de le supprimer, cela dit, nous avons connu un certain nombre de déceptions qui font que si nous ne nous opposerons pas ce texte, nous ne pourrons le voter telle quelle, c'est pourquoi nous nous abstiendrons pour 3, essentiellement premièrement le report, dans les faits, de la clause de revoyure au 30 juin 2023 alors que l'Assemblée avait voté le 31 janvier deuxièmement le fait que pour la possibilité de contrôle au plan international et je salue d'ailleurs la position qui a été celle de Monsieur le Ministre notre assemblée et choisit de restreindre les modalités du contrôle au test excluant la vaccination, ce qui pose un véritable problème alors que nous avons tellement milité les uns et les autres sur l'ardente nécessité de la vaccination, sur la question de l'article 2 bis, nous considérons qu'il a été introduit de manière artificielle, qu'il ne règle pas le problème qui est posé et qu'il aboutit à une sorte d'aporie de telle manière qu'une fois que la question ne se posera plus, elle est censée ne pas se poser, il ne s'agit pas de réintégration, comme le dit d'ailleurs, monsieur le rapporteur, toujours est-il que cela n'apporte rien de positif donc, mes chers collègues, pour ces raisons, nous nous abstiendrons dans l'espérance, que la commission mixte paritaire qui aura lieu demain permettra de nouvelles avancées qui nous.

Oui merci madame la présidente, monsieur me ministre monsieur le rapporteur, donc nous, nous nous apprêtons à à nous prononcer sur ce 11ème, texte de mesures sanitaires dans un contexte où je préfère le dire, le rapport de force entre Assemblée nationale et Sénat est désormais différent, je pense qu'il est nécessaire de le préciser, pour aujourd'hui et pour les textes à venir car je pense que cela a du sens, alors monsieur le rapporteur nous propose un texte réécrit qui est, qui est bien plus acceptable que la version du gouvernement mais d'une part, certaines mesures bien qu'améliorée perdure le passe sanitaire étant supprimé mais restant en suspens : si la situation empire variant d'un jeu dangereux émergents et système de santé saturé, particulièrement en outre-mer remplacé donc par un certificat sanitaire de voyage, d'autre part, nous, nous, nous nous interrogeons sur l'issue de la CMP, jusque-là, les sénateurs, ou plutôt la droite sénatoriale n'a pas eu gain de cause, ainsi, nous espérons que cette fois, et je l'ai dit dans mon intervention général Monsieur bah tiendra ses positions notamment sur ces réécriture des articles phares, hein, et de, pour l'heure, je veux le dire avec force en responsabilité parce que nous sommes des gens responsables des parlementaires responsable, nous ne pouvons voter un tel texte sans garantie ni sur les systèmes d'information, ni sur le droit d'initiative des élus ultramarins quant à la mise en oeuvre du certificat sanitaire de voyages, suite à la saturation des systèmes hospitaliers des territoires. Merci. Monsieur le président, Richard. Oui, Monsieur le Président, Retailleau. Merci madame la présidente, ça n'est pas le 1er texte sanitaire qu'on s'apprête à voter très majoritairement pour notre groupe, c'est le treizième mais c'est le premier. Qui fait l'objet d'un examen dans cet hémicycle, dans une nouvelle donne politique et parlementaire. Le Sénat comme à l'habitude. A fait son travail, faut-il rappeler que le texte qui nous est arrivé. était un moyen de texte amputé d'une grosse partie de sa consistance. Il est arrivé, amputé, il va repartir compléter. Et réécrit très profondément, je voudrais remercier la commission des Lois Philippe Bas notre excellent rapporteur du travail qu'ils ont fait tout au long de cette réécriture de cet examen, le Sénat a poursuivi sa ligne sa méthode habituelle, qui est une méthode d'exigence, l'exigence de clarté. Nous avons mis explicitement enfin. Au régime d'exception. Pour les états d'urgence sanitaire. Un régime et surtout une exigence aussi en matière de maîtrise de contrôle du Parlement, ça ne sera pas le gouvernement qui aura le bon vouloir de décider de réintégrer ou non les personnels soignants. Il y a un dispositif qui est créé exigences aussi en matière de maîtrise des frontières j'avais suffisamment à l'époque, pendant la première année, critiquer le gouvernement. De ce paradoxe puisque on ouvrait toutes grandes les frontières au moment où on replaçait devant le domicile des gens des frontières des petites frontières avec le confinement c'était incompréhensible et enfin une exigence aussi pour que le dispositif soit strictement proportionnée. Nous sommes toujours favorables à la vaccination, mais nous pensons qu'en matière de contamination le l'instrument le plus robuste, c'est le dépistage, c'est donc un un message, un message pour le gouvernement, qui devra compter sur avec le Sénat et c'est le retour du Parlement mais madame la présidente, permettez-moi de dire que dans le retour du Parlement, c'est aussi le l'affirmation d'un bicamérisme qui sera désormais plus équilibré. Merci monsieur le président, Richard. Madame la présidente, nous arrivons au terme d'un débat qui a été bien menée et dans lequel je salue en particulier : la volonté du gouvernement d'arriver à un texte répondant aux besoins, poursuivant les objectifs qu'il avait fixé au départ, mais tenant compte dans le dans le dialogue dans la délibération des apports de du Sénat dans sa diversité, puisque les votes que nous avons eu sur les différentes composantes du texte ont été parfois contrastées, il me semble donc le gouvernement et la majorité qui va s'exprimer ce soir en faveur de ce texte au Sénat ont largement contribué à aboutir à un texte responsable, un texte efficace et un texte qui peut devenir applicables dans les jours qui viennent, à l'issue de la commission mixte paritaire dans le bicamérisme, j'ai entendu parfois des allusions plus ou moins critiques à ce qui se passait à l'Assemblée nationale, il me semble que quand on veut vraiment légiférer vraiment faire la loi, on est amené à anticiper sur ce que sera aussi la préoccupation de l'autre assemblée pour arriver à à un accord équilibré, il me semble que c'est ce que nous avons fait le gouvernement il y a largement contribué, il me semble donc que nous sortions, nous sortons avec l'approbation qui va survenir de ce texte avec une bonne préparation de la future législation. Merci. Alors donc, je l'avais dit j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe, les républicains sur l'ensemble du texte, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos. Si, Si, alors voici le résultat du scrutin numéro 123 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence Nombre de votants : 342 Nombre de suffrages exprimés 222 pour l'adoption 189 contre 33, le Sénat a adopté. Mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance jeudi 21 juillet à 11 heures pour le projet de loi autorisant la ratification des protocoles du traité de l'Atlantique nord sur l'accession de la République de Finlande et du royaume de Suède, la séance est levée.